La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 26 octobre 2017 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Nelly Olin, qui fut sénateur du Val-d'Oise de 1995 à 2004. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,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 par l'inscription, sous réserve de sa transmission, du projet de loi de finances rectificative pour 2017. Acte est donné de cette demande. La commission des finances se réunira pour examiner le rapport le mercredi 8 novembre au matin. Le délai limite de dépôt des amendements sur ce texte pourrait être fixé au jeudi 9 novembre, à midi, et la réunion de la commission pour l'examen des amendements, au début d'après-midi. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Les Républicains, de la discussion de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage, présentée par M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues, en examen conjoint avec la proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé, présentée par M. Loïc Hervé et plusieurs de ses collègues.

Le texte que j'ai déposé et qui a été cosigné par nombre de mes collègues du groupe Les Républicains s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi Besson du 5 juillet 2000, qui est un texte équilibré, accordant à chacune des parties des droits et devoirs droit pour les gens du voyage d'être accueillis, dans le cadre d'un schéma d'accueil départemental, et, en contrepartie, devoir pour eux de respecter les clauses de ce schéma devoir pour les collectivités territoriales de réaliser les aires d'accueil inscrites dans le dispositif d'accueil départemental et, dans ce cas, droit d'attendre des pouvoirs publics l'évacuation des personnes et véhicules qui occupent illicitement un terrain. Or, aujourd'hui, cet équilibre entre droits et devoirs est rompu. Le cadre législatif de 2000 n'est plus adapté aux réalités de 2017. Les flux de gens du voyage sont de plus en plus nombreux et s'étalent sur une durée plus longue. Cette année, les premiers rassemblements en Haute-Savoie ont débuté au mois de février et perdurent encore à l'heure actuelle. Un certain nombre de personnes, peut-être en rupture avec la vie urbaine, choisissent ce mode de vie sans en partager la culture et viennent s'agréger aux voyageurs traditionnels. Les incidents sont de plus en plus fréquents et plus violents. Aux insultes s'ajoutent des agressions physiques envers les élus, qui veulent que la loi soit respectée, mais aussi envers les agriculteurs, les entrepreneurs, qui souhaitent protéger leur outil de travail. Des élus ont été frappés, dans le Nord comme en Haute-Savoie : c'est totalement inacceptable. Les maires sont désarmés, se sentent peu soutenus et sont véritablement exaspérés. Dans son bilan sur l'accueil des gens du voyage en Haute-Savoie, le préfet l'affirme clairement : « L'accueil des grands groupes dans le département doit désormais tenir compte de l'exaspération de nombreux élus locaux face à la multiplication des stationnements illicites. La population est excédée, elle ne comprend pas que, d'un côté, la loi s'applique avec sévérité lorsque l'on dépasse, ne serait-ce que d'une heure, la durée autorisée de stationnement en ville, et que, de l'autre, on fasse preuve de laxisme envers des personnes qui stationnent de façon totalement illicite plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sur des terrains publics ou privés, en toute impunité, procédant à des branchements sauvages pour s'alimenter en eau et en électricité et laissant ces terrains dans un état de dégradation inacceptable. Nos compatriotes reprochent alors à leur maire cette inaction ou ce laxisme. C'est injuste, car, dans la plupart des cas, il n'y a ni inaction ni laxisme. Simplement, les procédures et le cadre législatif actuels ne sont plus adaptés. Mme le procureur du tribunal de grande instance d'Annecy a déclaré très clairement devant les maires de Haute-Savoie réunis en congrès le 21octobre dernier : « En l'état actuel du droit, n'attendez rien de plus de l'autorité judiciaire. Mes chers collègues, la loi Besson n'est plus efficiente, elle doit être modifiée. C'est l'objet de ma proposition de loi et de celle de notre collègue Loïc Hervé.

Si nous voulons avancer, nous devons le faire dans un esprit de concorde, et non d'affrontement. Pour cela, il nous faut éviter deux écueils. Le premier serait de faire preuve d'un angélisme naïf et de nier la réalité

le préfet et la ministre de procéder à des évacuations rapides, tant la situation est intolérable. Le second écueil, c'est l'amalgame et la stigmatisation des gens du voyage. Ces situations problématiques sont le fait non de l'ensemble des voyageurs, mais d'une minorité d'entre eux qui bafoue nos lois et qui, de ce fait, porte préjudice à l'ensemble des communautés. Ma proposition de loi tend d'abord à responsabiliser et, si nécessaire, à sanctionner, car une sanction n'a de sens que si elle a été clairement expliquée. Mes chers collègues, sortons de ce débat d'un autre siècle qui voudrait opposer information, éducation et sanction. Au contraire, conjuguons-les : c'est le sens de ce texte, dont le premier volet clarifie le rôle de l'État et celui des collectivités territoriales. de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence obligatoire pour l'aménagement, l'entretien et la gestion des terrains d'accueil, sans en tirer les conséquences dans la loi Besson.

pour rappeler la compétence des EPCI en matière de création des aires et terrains. Cet article tend également à faciliter les efforts de mutualisation au sein d'un EPCI. Par souci de clarté, il exclut explicitement des schémas départementaux les EPCI ne comptant aucune commune de plus de 5 000 habitants, seuil fixé par la loi Besson.

à l'encontre des collectivités territoriales à l'heure où celles-ci doivent faire face à une baisse des dotations de l'État, comme l'a déploré la Cour des comptes, qui a estimé le coût moyen d'une aire d'accueil à 35 000 euros. L'article 3 tend à répondre aux problèmes rencontrés par les élus locaux. Il prévoit un mécanisme d'information afin de mieux anticiper les rassemblements et passages et confie au préfet le pouvoir de police lors de ces manifestations. Le chapitre II a trait à la modernisation des évacuations et stationnements illicites. Ses trois articles visent à améliorer l'efficacité des procédures, à renforcer les sanctions pénales, à interdire le phénomène des « sauts de puces » et à empêcher les personnes concernées d'aller s'installer à quelques mètres du terrain évacué, comme c'est souvent le cas actuellement. L'article 4, auquel j'associe notre collègue Jean-Pierre Grand, met fin à une interprétation erronée de la loi Besson figurant dans une réponse ministérielle du 31 octobre 2013. Il précise qu'une commune qui remplit ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage est en droit de demander l'évacuation des campements illicites, même si elle appartient à un EPCI qui ne respecte pas ses engagements. L'article 5 précise que la mise en demeure de quitter les lieux concerne la totalité du territoire de la commune ou de l'EPCI, afin, je le répète, d'empêcher les personnes concernées de s'installer à quelques mètres du collègues, je vous propose d'ajouter aux troubles à l'ordre public l'évacuation lorsque l'occupation illicite du terrain est de nature à entraver une activité économique ou agricole, y compris s'agissant des terrains en jachère. Je vous propose également deux mesures pour accélérer les procédures administratives : d'une part, réduire le délai d'exécution de la mise en demeure du préfet de vingt-quatre à six heures lorsque les mêmes personnes ont déjà indûment occupé le terrain de la commune ou d'une autre commune de l'EPCI au cours de l'année à quarante-huit heures au maximum le délai de recours contre la mise en demeure du préfet, alors qu'en l'état actuel il n'existe aucun délai uniforme pour ce recours suspensif. De plus, De plus, le préfet pourrait faire procéder à l'évacuation si un terrain d'accueil est disponible à moins de cinquante kilomètres. L'article 6 renforce les sanctions pénales. Il tend à doubler les peines encourues, en les portant à un an d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende. Il crée un mécanisme de pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par jour et par véhicule. Enfin, je vous propose de renforcer la saisie des véhicules et de permettre le transfert

Loïc Hervé et celles qui ont été introduites par la commission des lois, présidée par Philippe Bas, dont chacun connaît le sens de la mesure. Permettez-moi de saluer le travail rigoureux, méticuleux du rapporteur, Catherine Di Folco. son pragmatisme, sa sérénité ont permis d'enrichir considérablement ce texte. En effet, madame la ministre, mes chers collègues, c'est bien de la sérénité qu'attendent les élus, toujours en première ligne et dont je salue l'esprit de responsabilité. C'est aussi de la sérénité qu'attendent la majorité des gens du voyage, victime d'une minorité qui ne respecte pas nos lois. C'est enfin de la sérénité que réclame la population, qui sait que le « vivre ensemble » est l'ADN de la France, à condition que chacun respecte l'autre. Dans notre République, la loi doit énoncer clairement le cadre des droits et devoirs de chacun, car la liberté, fût-ce celle de circuler, s'arrête où commence celle de l'autre. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, il y aurait, dans notre pays, des sujets plus difficiles à aborder que d'autres ; si difficiles d'ailleurs que le législateur devrait être précautionneux, tant et si bien que l'abstention devrait prendrait le pas sur l'action. Assurément, c'est le cas du sujet de l'accueil des gens du voyage. Peut-être en est-il ainsi parce qu'il s'agit de la vie quotidienne de nos compatriotes, peut-être parce que notre rapport à cet accueil reste complexe, sans doute parce que nous craignons d'être nous-mêmes victimes de nos représentations et préjugés. D'emblée, je veux tordre le cou à une forme d'inversion des responsabilités. On nous explique que les torts seraient du côté des élus qui, ne respectant pas la loi Besson et les obligations du schéma départemental, seraient les responsables d'une situation dans laquelle ils se seraient eux-mêmes placés. Eh bien, il faut regarder la situation en face : dans nos départements, les élus, au travers de leurs communes, des syndicats compétents, des intercommunalités, ont, conformément au schéma départemental, engagé des investissements considérables dont ils assument aujourd'hui les charges et déficits de fonctionnement. Ce sont des choix difficiles qu'il leur faut assumer devant leurs concitoyens. Je parle en connaissance de cause, puisque, dans la communauté de communes dont je suis le président pour quelques heures encore, la construction de trente places d'accueil, il y a deux ans, a coûté la somme rondelette d'un million d'euros, hors foncier. En Haute-Savoie, territoire par territoire, nous sommes en conformité avec le schéma départemental ou en passe de l'être sur tous les sujets : aires d'accueil, aires de grand passage, aires de sédentarisation. La Haute-Savoie est un département de lacs et de montagne, un département dynamique et frontalier, un département accueillant et attractif, y compris pour les gens du voyage. Pourtant, chaque année, souvent dès le mois de février, comme l'a rappelé Jean-Claude Carle, de très nombreux stationnements illicites sont constatés sur tout le territoire, sur des parcelles agricoles, sur des tènements économiques, interrompant parfois l'activité des entreprises -cela a été le cas dans ma commune cette année année -, sur des équipements publics, en empêchant même la jouissance paisible par les associations et nos concitoyens. Si notre département est ouvert sur le monde et accueillant, ne nous leurrons pas : l'offre d'aires aménagées ne répondra jamais à une demande toujours croissante.

je précise d'ailleurs que c'est au travers d'un travail de fond avec les élus, mais aussi avec les acteurs de la justice, de l'éducation nationale ou de la sécurité, comme les gendarmes, que nous avons élaboré des propositions de nature à répondre concrètement aux difficultés suscitées par les stationnements illicites.

mais aussi aux élus locaux un moyen d'action concret et efficace. Aujourd'hui, nos concitoyens ont trop souvent le sentiment que ces acteurs sont de simples spectateurs de ces occupations illicites, dépourvus de tout moyen d'action ... Aujourd'hui, c'est la réalité de terrain qui nous appelle à légiférer de nouveau. Le texte résultant des travaux de la commission des lois dont nous allons débattre est issu de deux propositions de loi rédigées par mon collègue Jean-Claude Carle

C'est bien la réalité quotidienne vécue par les élus qui nous a alertés et poussés à regarder ce qui, dans la loi, pouvait être encore amélioré. Oui, au travers de nos propositions de loi, de nos prises de parole, ce sont de très nombreuses communes et leurs élus qui interpellent le Sénat et qui réclament une prise en compte de ce qu'ils vivent. Certains de ces élus sont présents en tribune cet après-midi pour écouter nos débats ; je les salue cordialement. Dans tout le pays, de nombreux maires, présidents d'intercommunalité ou de syndicat, de bonne volonté et respectueux de la loi, font face chaque année à des situations difficiles dans lesquelles cette même loi est ouvertement bafouée, comme le sont les droits des riverains, des dirigeants économiques, des agriculteurs, des collectivités, et ce des semaines durant, les dégradations se chiffrant souvent en dizaines de milliers d'euros d'argent tant privé que public.

stigmatisation ». Certains pensent qu'il faudrait complètement récrire la loi Besson. Ce n'est pas mon cas, et je ne crois pas utile de revenir sur les fondements de ce texte. En revanche, clarifier le rôle de l'État et celui des collectivités territoriales et des EPCI, améliorer l'information, moderniser les procédures d'évacuation des terrains occupés illicitement me paraît assurément indispensable, de même qu'adopter les mesures qui permettront de renforcer l'arsenal pénal et de rendre plus effectives les peines prononcées. Je tiens à remercier très sincèrement Mme le rapporteur, Catherine Di Folco, de son travail d'analyse, de synthèse et d'enrichissement. Chacune des mesures proposées a été pesée et consolidée juridiquement ; je m'en réjouis. Madame la ministre, vous êtes très bien informée des remontées du terrain. Vous avez d'ailleurs pris le temps de recevoir élus et agriculteurs de la Haute-Savoie à la fin du mois de juillet. Vous savez les difficultés suscitées par certains stationnements illicites des gens du voyage, vous savez que cette situation inquiète les élus, parfois même les épuise. Vous savez aussi que cette question pose problème au regard de notre pacte social. Madame la ministre, l'État de droit existe quand la loi votée par le Parlement est appliquée par l'administration et l'autorité judiciaire dans les décisions qu'elles prennent ou rendent. lors que la loi soit rédigée de manière à résoudre les troubles à l'ordre public ou les atteintes à la propriété privée. L'État de droit existe quand les décisions administratives ou judiciaires donnent lieu à une exécution rapide. Quand le sentiment d'impunité se répand, c'est la République qui s'affaiblit et c'est la force même de la loi qui en pâtit. Il y va de la crédibilité de l'État, du Parlement, de la justice, des élus locaux, de la police et de la gendarmerie.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la commission des lois a examiné conjointement la proposition de loi de M. Jean-Claude Carle tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage et la proposition de loi de M. Loïc Hervé visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé. En matière d'accueil, d'habitat et de stationnement des gens du voyage, notre droit se caractérise depuis bientôt trente ans par la recherche d'un équilibre entre droits et devoirs de chacun. Néanmoins, cet équilibre demeure précaire. Force est de constater que, d'un côté, les aires et terrains d'accueil destinés aux gens du voyage ne sont pas en nombre suffisant, notamment en raison du désengagement financier de l'État, ... Très bien ! ... qui ne finance plus depuis 2009 la réalisation des aires d'accueil et terrains familiaux, sauf pour les communes nouvellement inscrites au schéma départemental. départemental. Ainsi, les crédits de paiement inscrits à cette fin en loi de finances sont passés de 46 millions d'euros en 2008 à 5,3 millions d'euros dans le projet Quant à l'aide au fonctionnement, selon le rapport de 2017 de la Cour des comptes, la réforme de l'aide au logement temporaire à compter du 1 janvier 2015 a fait baisser les montants versés de 36,7 millions d'euros en 2014 à 32 millions d'euros en 2015. Toutefois, de gros progrès ont été réalisés ces dernières années. Selon un rapport du ministère du logement, en 2016, le nombre de places disponibles en aires permanentes d'accueil aménagées s'élevait à 26 873, soit un peu plus de 70 % du total des prescriptions des schémas départementaux. En revanche, le retard est plus important concernant les aires de grand passage : selon la Cour des comptes, 170 aires avaient avaient été réalisées au 1 janvier 2014, soit environ 50 % du total prescrit. Madame la ministre, les communes devant faire face depuis plusieurs années à de multiples charges supplémentaires sans compensation, à une diminution importante des dotations, je ne peux qu'inviter le Gouvernement à prendre l'initiative de rétablir le subventionnement par l'État des aires d'accueil et des terrains familiaux, pour donner aux communes les moyens d'exercer leur compétence. Par ailleurs, il convient de souligner que nombre d'aires et de terrains ont un taux de fréquentation relativement faible, aux alentours de 55 %. D'un autre côté, cela vient d'être précisé, les stationnements illicites perdurent, et auraient même tendance à se multiplier. Les élus locaux manquent de moyens pour faire cesser ces troubles. Il n'est pas question ici de mettre au ban de la société les gens du voyage, ... Absolument ! ... dont le mode de vie itinérant mérite respect et considération. Ils se sont vu reconnaître de longue date par la République le droit d'être accueillis sur le territoire des communes où ils viennent à s'établir. Lors des auditions, les représentants des associations de gens du voyage qui ont bien voulu répondre à notre invitation- certains ont refusé -ont déclaré que ceux-ci voulaient être traités comme tout citoyen français. Or, faut-il le rappeler, tout citoyen français a des droits et des devoirs : s'il ne respecte pas ces derniers, il encourt des sanctions. L'objet principal de ces deux propositions de loi est d'apporter des réponses concrètes aux problèmes posés par les installations illicites, en clarifiant le contenu et les modalités de mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage instauré par la loi du 5 juillet 2000, en assurant une meilleure préparation des grands passages, en facilitant l'évacuation des résidences mobiles irrégulièrement installées et en renforçant la répression pénale de ces comportements. La commission des lois a adopté vingt-quatre amendements visant à inclure dans la proposition de loi de M. Carle les principaux apports de la proposition de loi de M. Hervé, à améliorer ou compléter les dispositions proposées et à remédier à certaines difficultés juridiques. concerne le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, la commission a clarifié la répartition des rôles entre communes et EPCI dans sa mise en oeuvre. À l'article 1, elle a adopté un amendement de Mme Françoise Gatel et un autre de M. Jean-François Longeot tendant à apporter de nouvelles garanties aux élus locaux sur le contenu du schéma. À l'article 2, approuvant la suppression de la procédure de consignation de fonds à l'encontre des communes et EPCI défaillants, la commission, sans remettre en cause le pouvoir de substitution de l'État, a souhaité qu'il ne puisse s'exercer que six mois après la mise en demeure du préfet.

Toutefois, il ne lui a pas paru souhaitable de transférer au préfet le pouvoir de police municipale lors de ces événements. En effet, il est à craindre que ce transfert ne laisse les maires encore plus démunis en cas d'inaction du préfet et ne constitue un précédent fâcheux. Le droit en vigueur laisse ouverte la possibilité, pour le préfet, de se substituer au maire dans le cas où ce dernier n'aurait pas les moyens matériels d'assurer le maintien de l'ordre public. Concernant le pouvoir de police du stationnement des résidences mobiles, la loi du 5 juillet 2000 attribue au maire le pouvoir d'interdire le stationnement de ces dernières sur le territoire de la commune en dehors des aires et terrains aménagés à cet effet. À l'article 4, la commission a précisé les dispositions relatives à ce pouvoir de police spéciale et prévu de l'étendre aux maires des communes pourvues d'une aire d'accueil, même si l'EPCI auquel elles appartiennent n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations. Ce pouvoir de police spéciale est également étendu au président de l'EPCI, pour tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre les communes et leurs groupements. Concernant l'évacuation des campements illicites, malgré l'existence de différentes voies de droit, les élus locaux et les propriétaires des terrains peinent à obtenir une évacuation rapide. Cela tient notamment Cela tient notamment à l'insuffisance des moyens humains et matériels dont disposent les préfectures pour procéder à l'évacuation forcée d'office ou en exécution d'une décision de justice. À l'article 5, la commission a entendu accélérer la mise en oeuvre de la procédure d'évacuation d'office des résidences mobiles irrégulièrement stationnées en limitant le délai de recours contre la mise en demeure du préfet à et en fixant à vingt-quatre heures le délai d'exécution de la mise en demeure d'évacuer en cas de nouveau stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l'EPCI au cours de la même année. Afin de répondre aux préoccupations légitimes de nombreux élus locaux, la commission a adopté un nouveau cas de mise en demeure, en plus du trouble à l'ordre public. nouveau cas met en balance la liberté d'aller et venir des gens du voyage avec d'autres principes d'égale valeur constitutionnelle : le droit de propriété, la liberté d'aller et venir des autres habitants, la liberté du commerce et de l'industrie et la continuité du service public. La commission a également facilité le recours aux procédures juridictionnelles de droit commun que sont le référé administratif, le référé civil et la requête civile. Cette dernière procédure, non contradictoire, est particulièrement adaptée dans l'hypothèse- fréquente -où il est impossible d'obtenir l'identité des occupants sans titre. Concernant la répression pénale des occupations illicites, la commission a donné un avis favorable aux amendements de M. Hervé visant à renforcer le dispositif répressif. Cependant, la répression pénale ne peut avoir un effet dissuasif que si elle est effectivement mise en application- M. Hervé y a fortement insisté, et je partage son point de vue. Or ce n'est souvent pas le cas, faute de moyens, mais aussi de volonté de la part des procureurs de la République. L'article 6 modifie l'article 322-4-1 du code pénal relatif au délit d'occupation sans titre d'un terrain : il prévoit de doubler les peines encourues, qui seraient portées à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. également le transfert des véhicules destinés à l'habitation sur tout aire ou terrain aménagé à cet effet dans le ressort du département. Cet article instaure enfin une amende forfaitaire délictuelle. L'article 7 renforce les sanctions pénales en cas de destructions, dégradations ou détériorations du bien d'autrui. L'article 8 crée un délit d'occupation habituelle sans titre d'un terrain : au moins quatre contraventions sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois caractérisent l'habitude. L'article 9 permet l'application de la peine complémentaire d'interdiction de séjour en cas d'infraction d'occupation sans titre d'un terrain. L'article 10 prévoit l'application outre-mer des dispositions modifiant le code pénal. texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Un dernier élément contenu dans la proposition de loi de M. Hervé n'a pu être retenu car il relève du domaine réglementaire. Il s'agit de la présence obligatoire d'un représentant du directeur académique des services de l'éducation nationale au sein de la commission départementale consultative associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, afin de « mieux prendre en compte les besoins éducatifs des enfants, et de définir des actions éducatives et sociales destinées aux gens du voyage ». Ce sujet est effectivement très important : les enfants des gens du voyage sont soumis, comme les autres, à l'obligation scolaire. Or leur taux de scolarisation reste faible 70 % au niveau élémentaire, et de seulement 5 % au niveau du collège. Bien que des mesures aient été prises pour assurer le respect de l'obligation scolaire, il serait intéressant de faire un état des lieux de la scolarisation des enfants du voyage, afin d'identifier les difficultés qui subsistent et d'y apporter les réponses nécessaires. Madame la ministre, il conviendrait de veiller à ce que les services de l'éducation nationale soient systématiquement associés à la définition des politiques publiques en matière d'accueil, d'accompagnement social et éducatif des gens du voyage. Très bien ! La parole est

de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute Assemblée a souhaité remettre à l'ordre du jour la révision du cadre juridique applicable aux conditions d'accueil et d'habitat des gens du voyage qui résulte de la loi du 5 juillet 2000, dite « loi Besson ». Ce cadre avait fait l'objet de modifications substantielles au travers des lois territoriales de 2014 et de 2015, qui ont transféré la compétence aux métropoles et aux intercommunalités, et surtout au travers de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté adoptée sur l'initiative des députés Dominique Raimbourg et Bruno Le Roux. Je ne reviendrai pas sur le contenu des deux propositions de loi, qui ont été très précisément présentées par leurs auteurs, ni sur le contenu du texte résultant des délibérations de votre commission des lois, dont je veux saluer le travail, en particulier celui de son rapporteur, Mme Catherine Di Folco. Moins d'une année après l'entrée en vigueur de la loi Égalité et citoyenneté, fallait-il remettre sur le métier ces dispositions législatives, dont certaines n'ont pu encore faire l'objet d'une évaluation exhaustive de la part des ministères concernés ?

Ainsi, au cours de l'année 2017, le département de Haute-Savoie a été confronté à des installations illicites ayant affecté des terrains agricoles ou des zones industrielles, et donc l'activité économique à proximité de zones d'habitat. Ces situations provoquent des tensions parfois très vives avec les élus, les agriculteurs, les chefs d'entreprise et les riverains. De tels incidents, d'ailleurs non limités à ce seul territoire et qui sont souvent le fait de quelques groupes isolés, contribuent à l'évidence à créer un climat délétère. Ce climat participe, du reste, de l'amalgame que peut faire la population entre les auteurs de ces pratiques et la grande majorité des gens du voyage, dont l'installation sur les aires d'accueil n'engendre pas de troubles.

Ainsi, selon le dernier bilan établi par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, à la fin de l'année 2016, le nombre de places disponibles en aires permanentes d'accueil aménagées s'élevait à 26 755, soit

quelque progrès à faire concernant les terrains familiaux. Par ailleurs, comme le relève la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour l'année 2017, le nombre de places créées dans des aires d'accueil continue à progresser

Se pose bien entendu également la question de l'acceptation par les riverains de l'implantation de ces aires. La Cour des comptes relève enfin une tendance à l'« ancrage territorial territorial » des gens du voyage, qui conduit à une occupation quasiment permanente de certaines aires d'accueil, voire d'aires de grand passage, certaines faisant même l'objet d'une appropriation totale par des groupes familiaux.

Il nous appartient à tous collectivement, Gouvernement, administration, élus nationaux et locaux, de donner aux gens du voyage les moyens de vivre selon la manière qu'ils ont choisie. C'est tout l'objet et le sens de la loi du 5 juillet 2000, dont l'application doit être garantie, encouragée, accompagnée. Toutefois, ce mode de vie doit bien entendu s'exercer dans le respect des lois de la République, et le Gouvernement sera sur ce point très vigilant. Ce constat étant posé, est-il nécessaire de changer la loi ? Sûrement, sur certains aspects. Ainsi, il est clair que le transfert des compétences « aménagement, entretien et gestion des aires et terrains destinés aux gens du voyage » aux métropoles au travers de la loi MAPTAM,

de la loi du 5 juillet 2000. Il en résulte ce paradoxe, que vous êtes nombreux à souligner, que si les EPCI sont désormais compétents en la matière, les obligations découlant des schémas départementaux continuent à reposer sur les communes, alors même qu'elles sont dépourvues de moyens juridiques d'agir, en vertu du principe d'exclusivité des compétences transférées. Eh oui ! De ce point de vue, les réponses juridiques apportées par le texte élaboré par la commission des lois sont intéressantes et constituent une solide base de départ. De même, la commission des lois propose de donner un fondement légal à la procédure d'information préalable des communes et EPCI et de la formaliser, en vue d'organiser les grands rassemblements et, surtout, les grands passages qui les précèdent. Ces importants mouvements de groupes de gens du voyage, souvent composés de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de véhicules, font l'objet d'une attention toute particulière de la part des services de l'État, qui les préparent avec le plus grand soin, en liaison avec les collectivités concernées. Cette procédure, définie dans une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 10 avril 2017, s'appuie sur les principes de programmation des occupations successives des terrains pour prévenir les occupations illicites et de définition de conventions d'occupation cosignées par les collectivités et les représentants des associations. Ces conventions fixent, aussi précisément que possible, les conditions et délais de stationnement et permettent une responsabilisation des acteurs. Une telle formalisation, pour faiblement normative qu'elle puisse paraître, constitue également une base de réflexion intéressante. J'appelle néanmoins votre attention sur le fait qu'elle nous expose à un risque de non-application, dans la mesure où les arrivées de groupes sont parfois inopinées et en décalage avec les prévisions, les organisateurs n'ayant pas toujours les moyens et l'autorité nécessaires pour faire respecter la planification. En revanche, le Gouvernement ne saurait approuver les dispositions du texte soumis à votre délibération qui seraient de nature à affaiblir les obligations résultant des schémas pour les communes ou qui reviennent sur les outils dont dispose l'État pour les faire respecter.

aux collectivités qui auraient des projets de création d'aires d'accueil de solliciter un concours, au titre de la DETR, auprès des services de l'État. C'est un voeu pieux ! Par ailleurs, le Gouvernement est prêt à considérer les propositions visant à permettre de mieux lutter contre les occupations illégales de terrains. Je peux ainsi comprendre la réflexion introduite par la proposition de loi sur l'accès au pouvoir de police spéciale pour les communes ayant rempli leurs obligations, qui est aujourd'hui conditionné au respect par l'EPCI dans son ensemble de ses obligations. Je peux comprendre que de telles dispositions suscitent l'incompréhension des élus locaux qui, bien qu'ayant parfaitement respecté la loi, ne peuvent prescrire l'interdiction du ne peuvent prescrire l'interdiction du stationnement en dehors des aires réservées à cet effet. De même, le Gouvernement considère que l'application de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle au délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain en vue d'y établir une habitation constitue une piste intéressante pour améliorer la lutte contre les installations illicites. Le Gouvernement ne saurait en revanche approuver les dispositions de la proposition de loi dont la constitutionnalité apparaît fragile, à l'instar des mesures contenues à l'article 5,

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, je souhaiterais tout d'abord remercier la commission des lois et son président de s'être saisis des propositions de loi déposées par Loïc Hervé et Jean-Claude Carle.

à l'impuissance des élus locaux à gérer des situations de troubles. Je veux aussi saluer l'excellent travail accompli par notre collègue rapporteur Catherine Di Folco sur une thématique complexe et toujours délicate à traiter.

Afin de répondre au devoir d'accueil des gens du voyage et de mettre fin aux campements sauvages, la loi de 1990 avait prévu la réalisation d'aires d'accueil sur tout le territoire national.

Pour autant, nous le savons, cette procédure n'est applicable que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. Elle s'avère difficile à mettre en Si les procédures d'expulsion sont bien mises en oeuvre, les délais d'application sont très longs. Qui plus est, une fois expulsées, certaines communautés se réinstallent à quelques kilomètres, dans une autre commune, et la procédure d'expulsion doit alors être réengagée Ainsi, le dispositif juridique censé permettre aux élus de répondre à la question de l'accueil des gens du voyage se caractérise par sa grande complexité, laissant, trop souvent, les maires totalement démunis. Ces situations engendrent des dégradations dans les lieux occupés, des altercations parfois violentes, entre les gens du voyage et les habitants. Elles débouchent souvent sur des conditions d'accueil déplorables pour les gens du voyage, installés sur des terrains inadaptés. La présente proposition de loi, issue des propositions de loi déposées par Loïc Hervé et Jean-Claude Carle, vient utilement répondre aux difficultés rencontrées sur le terrain, en premier lieu à celles qui sont liées à l'installation illégale de gens du voyage sur des terrains publics ou privés. Je pense en particulier

Je pense également aux dispositions visant à remédier à une injustice subie par les maires s'étant acquittés de leurs obligations et ne pouvant faire usage de leur pouvoir de police en cas d'occupation illicite, dans l'hypothèse d'un manque d'emplacements sur le territoire intercommunal.

Pour autant, rappelons que la Cour des comptes a estimé, en 2012, que le coût moyen de réalisation d'une place en aire d'accueil est de 35 000 euros, auquel il convient d'ajouter les coûts de gestion et d'entretien de ces espaces. C'est pourquoi, dans un contexte de grande frugalité

l'exclusion du schéma départemental des groupements de communes qui ne comptent aucune commune de plus de 5 000 habitants va, me semble-t-il, dans le bon sens. Par ailleurs,

par la commission des lois de mon amendement visant à prendre en compte le taux d'occupation moyen des aires et terrains existants dans un même secteur géographique d'implantation pour mieux apprécier la pertinence de la

Le groupe Union Centriste votera donc cette proposition de loi, respectueuse de la citoyenneté des gens du voyage et du du devoir d'accueil des collectivités territoriales. Elle est aussi impérieusement nécessaire pour donner aux élus locaux les moyens indispensables à l'exercice des responsabilités que la loi leur a confiées. La parole

Comment ne pas l'être en effet lorsque nous sommes appelés à nous positionner sur un ensemble de mesures qui remettent en cause un dispositif concerté et équilibré, inscrit il y a dix mois à peine au sein de la loi Égalité et citoyenneté ?

et a fait l'objet d'un grand nombre de dispositions législatives et réglementaires depuis plus d'une trentaine d'années. Je tiens, à ce sujet, à rendre hommage aux élus locaux, qui, dans l'exercice de leurs missions toujours plus nombreuses au service de nos concitoyens, démontrent chaque jour à quel point leur action est essentielle, en particulier en matière d'aménagement du territoire et d'accueil de toutes les populations. C'est justement dans cet esprit qu'a été introduite en janvier dernier dans la loi une réforme concertée, discutée et équilibrée de la loi Besson du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La loi Égalité a ainsi précisé le contenu et les conditions d'élaboration des schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage, et a renforcé les dispositifs de mise en demeure et d'évacuation forcée en apportant trois améliorations au dispositif de la loi Besson, qui permet au maire d'interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées. Premièrement, elle permet de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir commis un premier stationnement illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain situé à proximité. Deuxièmement, elle réduit le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises en demeure. Troisièmement, elle elle clarifie le cas des terrains affectés à une activité à caractère économique. Dans le même temps, et dans un esprit de juste reconnaissance des droits et des devoirs de chacun, la loi

Entendons-nous bien : nous sommes, tout autant que les auteurs de ce texte, conscients des difficultés qui peuvent être rencontrées par les élus locaux en matière d'accueil des gens du voyage. Mais nous considérons que c'est précisément en rappelant et en faisant respecter les droits et les devoirs de chacune des parties prenantes que les choses pourront se trouver facilitées,

Quelle est l'utilité réelle d'une telle proposition de loi, qui revient sur des dispositions qui n'ont pas encore eu le temps d'être mises en oeuvre, et donc de faire leurs preuves, sauf à vouloir obtenir un effet d'affichage ?

l'immense majorité des élus des collectivités locales, ceux qui savent pertinemment qu'ils ne pourront remédier à des situations d'occupation illégale que si eux-mêmes

au 1 janvier 2014, 170 aires avaient été réalisées sur les 348 prescrites dans les schémas départementaux et, à ce jour, seuls 18 départements respectent leurs obligations en la matière ... Rappel des droits et des devoirs de chacun, respect des dispositions récemment votées par la représentation nationale, confiance dans les élus locaux et intercommunaux : autant de principes qui seraient battus en brèche si la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui était adoptée par la Haute Assemblée.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, de nombreux maires subissent chaque année des occupations illicites de terrains par des gens du voyage

Ils sont totalement désemparés lorsqu'ils voient que les lois de la République ne sont pas respectées. Une telle situation est inacceptable ! Qui peut la nier aujourd'hui ? Quel sénateur, quelle que soit la famille politique à laquelle il appartient, peut affirmer qu'il n'a jamais été alerté par des élus de son département sur les désordres qu'engendrent les occupations illicites, sur les intimidations à l'égard des représentants de l'ordre public et de la population, sur les destructions, les dégradations ou les détériorations de biens publics ou privés Mes chers collègues, si nous voulons pacifier les relations entre les Français sédentaires et les gens du voyage, il faut donc donner plus de droits aux communes et plus de moyens juridiques à leurs

les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont dû engager de lourds investissements afin d'accueillir les gens du voyage. Ainsi, toutes les communes de plus de 5 000 habitants ont été placées dans l'obligation de mettre en place une aire permanente d'accueil. En outre, en application des prescriptions du schéma départemental, elles ont pu se voir imposer la mise en place d'une aire de grand passage. Pour information, en 2018, la métropole européenne de Lille, dont je suis élu, a pour objectif de créer 310 places d'aire permanente d'accueil et 200 places d'aire de grand passage, ce qui représente une dépense de plus de 4 millions d'euros en investissement et de 3 millions d'euros en fonctionnement, pour une recette globale de 1 million d'euros. Quand on sait que ces dépenses d'investissement accroissent les besoins de financement des collectivités, on peut s'interroger sur leur réalisation si l'article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques est voté et appliqué dans sa rédaction actuelle, sachant que les collectivités territoriales respectent déjà des règles financières strictes en matière d'équilibre budgétaire. Mais nous aurons l'occasion d'en parler lors d'un prochain débat, mes chers collègues. Les deux propositions de loi réunies en une seule par la commission des lois qui nous occupent tendent à permettre un meilleur équilibre, en matière de droits et de devoirs, entre les gens du voyage et ceux qui les accueillent. Leurs dispositions prévoient tout d'abord de clarifier le rôle de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage de moderniser les procédures d'évacuation des stationnements illicites ; enfin de renforcer et de rendre plus effectives les sanctions en cas d'installation illégale en réunion sur un terrain public ou privé. Dans le texte issu des travaux de la commission, l'article 7, s'inspirant de l'article 3 de la proposition de loi de notre collègue Loïc Hervé, vise à créer, à l'article 322-3 du code pénal, une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui prévu à l'article 322-1 du code pénal. Ainsi, les peines encourues seraient de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende en cas de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui à l'occasion d'une installation illicite. Ces peines pourraient être portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique

je suis favorable à ces dispositions. Renforcer les sanctions pénales, c'est envoyer un signal fort aux magistrats, pour leur dire que les infractions commises par les gens du voyage doivent être sanctionnées. Sans sanction, il n'y a pas de dissuasion, et l'on consacre alors une impunité réservée à certains citoyens ! Je voudrais également dire un mot sur le schéma d'accueil des gens du voyage. Actuellement, le dispositif d'accueil est défini à l'échelle départementale. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil départemental. On peut regretter l'absence de concertation ou de discussion globale entre départements limitrophes sur ce sujet. Je pense que la mise en place d'un schéma interdépartemental d'accueil des gens du voyage constituerait une solution pertinente. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur les délais de procédure en matière d'évacuation en cas d'occupation illicite. Je regrette que les délais de la procédure administrative soient plus longs qu'en matière civile, tout comme je regrette que le parquet renonce trop souvent à poursuivre en cas de destruction, détérioration ou dégradation de biens ... Pour conclure, ce texte répond aux attentes des élus locaux, qui sont confrontés tous les ans au déséquilibre entre les droits et les devoirs des gens du voyage et ceux des collectivités.

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, une fois de plus, le législateur se penche sur la question de l'accueil des gens du voyage, qui, régulièrement, plonge dans le désarroi les maires de nos communes et nos concitoyens. Car, face à cette question, l'État, comme souvent, ne prend pas ses responsabilités. Il transfère à l'échelon local des compétences et lui laisse sur les bras la charge financière des installations, en ayant le toupet d'exiger la réalisation de toujours plus d'aires d'accueil tout en diminuant sans cesse les subventions qu'il alloue en la matière. Rappelons tout de même que le coût de réalisation d'une place d'aire d'accueil est de 35 000 euros. Pour les plus grandes aires, cela peut représenter plusieurs millions d'euros ! On exige des installations qui sont boudées par les bénéficiaires eux-mêmes, s'installant trop souvent où bon leur semble. Ainsi, dans la région de Toulouse, deux aires de grand passage ouvertes l'été dernier n'ont été utilisées que par trois groupes, autres préférant s'installer ailleurs. Alors, plutôt que de brandir des menaces fiscales contre des communes qui font, la plupart du temps, de gros efforts financiers, l'État devrait faire régner l'ordre et la sécurité. Les occupations illicites sont innombrables et provoquent des tensions entre « accueillants » et « accueillis », voire des affrontements avec la police, comme cela a été encore le cas le 26 octobre dernier. Le blocage de l'autoroute A1 au mois d'août 2015 est également dans toutes les mémoires. Les gens du voyage sont des citoyens français et, comme cela a été opportunément rappelé, ils ont des droits, mais aussi des devoirs. Or, si l'État exige toujours plus d'aires d'accueil, l'expérience montre que, dans beaucoup trop de cas, ces communautés n'ont que faire des terrains qui leur sont préparés et s'installent en toute illégalité sur des terrains privés ou communaux. Très souvent, ces terrains sont laissés par la suite à l'abandon dans un état pitoyable, comme cela a été encore le cas voilà quelques mois dans le 11 arrondissement de Marseille, où un terrain de sport a été totalement dévasté, et comme c'est le cas chaque année lors du traditionnel rassemblement des Saintes-Maries-de-la-Mer. Je le dis sans haine, mais avec fermeté : il faut que les communautés de gens du voyage cessent de se croire partout chez elles. Les maires ne doivent pas être les seuls à respecter la loi Plusieurs éléments positifs apparaissent cependant dans ce texte : le caractère facultatif, dans certains schémas départementaux, de la réalisation d'aires d'accueil de faible dimension sur le territoire de communautés de communes rurales qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune de plus de 5 000 habitants ; la conservation par le maire de son pouvoir de police municipale ; l'accélération des procédures administratives d'évacuation des stationnements illicites ; enfin, le renforcement des sanctions pénales en cas d'occupation illicite d'un terrain.

Comme dans beaucoup d'autres domaines, il faudrait commencer par appliquer la loi existante. Face aux installations anarchiques des gens du voyage, le fond du problème, c'est un État lâche, volontairement impuissant à lutter contre une violation de la loi et du droit de propriété. Que des moyens soient donnés aux maires ainsi qu'aux forces de l'ordre afin que la loi, rien que la loi, mais toute la loi, soit appliquée ! L'accueil des gens du voyage ne pourra qu'en être mieux assuré et mieux accepté. La parole est à M. Yvon Collin. Madame la

les questions abordées par les deux propositions de loi de nos collègues Loïc Hervé et Jean-Claude Carle sont éminemment sensibles et hautement clivantes. S'affrontent, parfois violemment, la liberté d'aller et venir des uns et le droit de propriété des autres, l'aspiration à la tranquillité des riverains et les atteintes à l'ordre public. Disons-le d'emblée, la République ne saurait faire de distinction entre ses citoyens autres que celles qui sont fondées sur le mérite. Elle l'a pourtant fait jusqu'à très récemment au détriment des gens du voyage, les soumettant à un statut administratif exorbitant du droit commun et à d'importantes limitations de leurs libertés publiques. Cette même République ne saurait davantage accepter qu'une partie de la population se détourne de l'application de la loi. Je connais, comme tous ceux qui ont exercé des fonctions exécutives locales, les implications sur le terrain, dans nos collectivités, de l'accueil des gens du voyage. Nous avons tous en tête des exemples de bonne cohabitation entre gens du voyage et riverains ou,, des cas d'occupation illicite et répétée de propriétés publiques ou privées. Certains élus se sentent aujourd'hui désarmés, voire abandonnés par l'État et ses services, lorsqu'ils se retrouvent confrontés à des occupations illégales et à des dégradations d'ouvrages publics. Mais il est tout aussi Mais il est tout aussi inacceptable que certaines communes s'affranchissent de leurs obligations légales en termes de réalisation d'aires d'accueil. Ceux qui, comme moi, ont un peu d'expérience se souviennent de la loi Besson de 2000, et des retouches qui y ont été apportées en 2003 et en 2007.

Il y a de cela quelques mois à peine, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, nous avons eu à examiner plusieurs articles qui abordaient plus globalement l'épineuse question de la place des gens du voyage dans notre société. Cette loi Égalité et citoyenneté a été publiée au à la fin de janvier 2017. À ce jour, toutes ses dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur,

Sur certaines travées, d'aucuns parmi nos collègues estiment que la loi Égalité et citoyenneté ne va pas assez loin. Je suis, pour ma part, plutôt enclin à laisser à la nouvelle loi le temps de s'appliquer. Nous pourrons, ultérieurement, procéder à son évaluation- je pense, par exemple, au mécanisme de consignation -et proposer éventuellement des améliorations. En effet, nous le savons, en matière d'accueil des gens du voyage, le principal écueil réside dans les difficultés à faire appliquer la loi, toute la loi. En outre, les lois de 2000 et de 2017 reposent sur un équilibre, imparfait sans doute, mais qui prévoit le respect, par chacun, de ses droits et de ses devoirs : par les collectivités locales,

l'État, enfin, qui doit être le garant de cet équilibre et affirmer la solidarité nationale. Or, il n'en va pas de même du texte que nous examinons aujourd'hui. Celui-ci n'est pas sans rappeler la proposition de loi de Pierre Hérisson, dont nous avions entamé l'examen fin 2013 et début 2014, opportunément quelques mois avant les élections municipales

Certaines des dispositions contenues dans le chapitre I, notamment celles visant à mieux prendre en compte les nouvelles compétences des intercommunalités, peuvent recueillir notre assentiment. Il n'en va pas de même des articles qui remettent en cause les grands équilibres que j'évoquais. Je pense, notamment, à ceux qui prévoient d'alourdir les sanctions pénales- nous aurons l'occasion d'y revenir Nous abordons donc l'examen de ce texte en étant pleinement conscients des problématiques qu'il soulève et convaincus qu'elles doivent être abordées avec responsabilité et dans un esprit de concorde. Quant au vote final des membres du RDSE, il dépendra, vous l'aurez compris, du sort réservé aux amendements

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, chers Jean-Claude Carle et Loïc Hervé, quelle quête que celle de l'équilibre entre mode de vie des itinérants et respect de la réglementation, particulièrement, du stationnement des résidences mobiles ! Le législateur s'y attache régulièrement et la présente proposition de loi s'inscrit dans cette démarche. Les plus hautes juridictions s'y sont engagées également. Le Conseil d'État, en 1983, avait eu l'occasion de consacrer le droit pour les gens du voyage d'être accueillis sur le territoire des communes où ils viennent s'établir et de reconnaître leurs véhicules comme des domiciles dont l'inviolabilité est constitutionnellement garantie. Le Conseil constitutionnel a pu rappeler, le 9 juillet 2010, que la liberté d'aller et venir constituait également une liberté constitutionnellement garantie.

Les schémas d'accueil prévus par la loi Besson se concrétisent peu à peu. Dix-sept départements ont déjà atteint leurs objectifs. La Seine-et-Marne, elle aussi attractive, pour d'autres raisons que la Haute-Savoie,

La dernière raison avancée par la Cour des comptes est la faible mobilité des gens du voyage due à la scolarisation des enfants- celle-ci reste au demeurant bien trop faible -, à leur plus grande précarité financière, à la fragilité juridique de leur installation et à l'absence de garantie de retrouver une place sur leur terrain d'élection.

Il nous semble ainsi difficile d'exclure du dispositif 45 % des intercommunalités de la Nation, celles qui ne comptent aucune commune de plus de 5 000 habitants, comme le prévoit l'article 1. Le caractère dissuasif du doublement des peines encourues prévues à l'article 322-4-1 du code pénal en cas d'occupation illicite peine, hélas, à convaincre quand on sait que soixante condamnations seulement ont été prononcées en 2016 pour ce délit, dont cinq à des peines d'emprisonnement ferme.

L'article 6, qui vise à étendre la confiscation des véhicules prévue par l'article 322-4-1 du code pénal à ceux destinés à l'habitation paraît difficilement conciliable avec le principe constitutionnel d'inviolabilité du domicile et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 8, 8, qui prévoit la création d'un délit de fraude d'habitude d'installation sur le terrain d'autrui, soulève quelques difficultés d'application, sans pour autant être dépourvu de fondement. Cela étant, nous soutenons

la création, à l'article 3, d'un mécanisme d'information obligatoire pour faciliter l'organisation de l'accueil des gens du voyage lors des grands passages et des grands rassemblements. l'article 4, qui prévoit notamment d'étendre aux maires des communes dotées d'une aire d'accueil conformément aux prescriptions du schéma départemental le pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles même si l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. Enfin, bien évidemment,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'accueil des gens du voyage est un véritable casse-tête et une source de conflits et de difficultés permanente pour les élus locaux

À ce jour, trois textes règlent les conditions d'accueil des gens du voyage par les collectivités : les lois Besson, MAPTAM et NOTRe, auxquelles s'est ajoutée la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Comme vous le savez, c'est la loi Besson du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage qui a posé les bases de la législation, en attribuant la compétence en matière d'aires d'accueil des gens du voyage aux collectivités territoriales et en inscrivant dans la loi l'obligation, pour les communes de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, de créer des aires d'accueil. Les lois MAPTAM et NOTRe attribueront par contre aux EPCI, en tant que compétence obligatoire, celle de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion de ces aires d'accueil.

ne manifestant pas un grand enthousiasme pour faire évacuer par la force publique les contrevenants qui s'installent là où bon leur semble, parfois même quand existe une aire d'accueil réglementaire sur le territoire de la commune. Ces retards, voire ces absences de réaction de la part des pouvoirs publics sont source d'incompréhension pour les élus, si ce n'est de rejet par le voisinage, qui en vient à se demander s'il n'y a pas deux catégories de citoyens : ceux que l'on sanctionne quand ils ne respectent pas la loi et ceux qui peuvent se le permettre en toute impunité. Notre sentiment est que nous ne sortirons de l'impasse qu'en faisant respecter la loi Besson par les uns et par les autres les collectivités en facilitant la réalisation des aires d'accueil, par les gens du voyage en facilitant la police des grands rassemblements ainsi que l'évacuation des terrains occupés illégalement dans les EPCI respectant la loi Besson et en renforçant les sanctions pénales en cas d'occupation illicite d'un terrain. Afin de faciliter terrain. Afin de faciliter la mise en oeuvre des schémas d'accueil, outre le rétablissement des financements de l'État- on peut toujours espérer ... -, il convient de clarifier la réglementation existante.

Par souci de cohérence, notre deuxième amendement tend à rétablir la consignation des fonds prévue par la loi Égalité et citoyenneté à l'encontre des collectivités qui ne respecteraient pas le schéma départemental d'accueil. Certaines n'ont absolument aucune envie de le faire

Mais si nous souscrivons aux dispositions qui visent à répondre à la situation, nous refusons celles qui sont inutilement répressives, et donc inefficaces. À quoi bon durcir les sanctions, multiplier les procédures expéditives quand on n'est pas capable d'appliquer celles qui existent, faute de volonté Quand vous aurez saisi les véhicules servant d'habitations, ce qu'exclut actuellement le code pénal, que ferez-vous des gens qui les occupent ? de retirer le permis de conduire à ceux qui contreviennent à la législation relative aux gens du voyage, elle n'aboutira, selon moi, qu'à l'augmentation du nombre de conducteurs sans permis,

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, le texte de loi qui nous préoccupe aujourd'hui est hautement attendu par de nombreux élus, notamment en Haute-Savoie. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si les trois sénateurs de la Haute-Savoie et ceux qui les ont précédés ont, tour à tour, déposé des questions orales ou écrites, rédigé des propositions de loi et interpellé, comme je le fais depuis trois ans, les différents ministres de l'intérieur qui se sont succédé. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à ma demande de nous recevoir au ministère de l'intérieur avec l'ensemble des acteurs concernés par la thématique des gens du voyage. Vous avez pu constater que la situation sur le terrain était préoccupante et que nous sommes assis sur une véritable poudrière, qui peut s'embraser à tout moment, d'un côté comme de l'autre. Afin de clarifier mes propos, je voudrais apporter quelques précisions. Tout d'abord, nous devons différencier les gens du voyage qui respectent les règles et représentent une très large majorité de ceux qui, au contraire, se comportent comme des délinquants et ne respectent pas les lois de la République et les arrêtés des communes ou des EPCI. maire d'une commune rurale de 1 500 habitants de 2008 à 2016, et pas une année ne s'est écoulée sans que je sois concerné par des installations illicites, ce qui a été le cas de nombreux maires cette année encore. Je connais donc bien le sujet, et il est important que je puisse relayer auprès de vous de façon factuelle le quotidien de ces élus de terrain, que comprend forcément moins bien l'administration.

Madame la ministre, les élus et les services de l'État s'investissent dans leurs missions. Les élus de mon territoire respectent leurs obligations légales, décidées dans le cadre du schéma départemental des gens du voyage. En effet, mon département dispose à ce jour de 16 aires d'accueil offrant une capacité de 488 places. Avec l'ouverture de l'aire de Reignier, l'ensemble du département est en conformité avec le schéma 2011-2017 concernant les aires d'accueil et de grands passages. Malgré cela, certains groupes semblent s'affranchir de droits fondamentaux, tels que le droit de propriété, qui est régulièrement bafoué. Concernant les petits groupes de gens du voyage, les troubles générés par les occupations illicites ont été particulièrement forts cette année en Haute-Savoie : 57 communes du département en ont subi au moins une et 103 demandes d'arrêtés de mise en demeure ont été formulées depuis le début de l'année, contre 89 en 2016- plus de 70 % sont le fait de deux familles. Concernant les grands passages, certains groupes se sont imposés, dans le département, par le nombre et la force, bien qu'un refus de séjour leur ait été notifié en début d'année, puis réitéré lorsqu'ils se sont annoncés la veille pour le lendemain. D'autres groupes arrivent aussi à leur convenance, méconnaissant les dates officielles de réservation. Les élus locaux n'en peuvent plus de passer des jours et des nuits à gérer les installations illicites, à subir invectives, menaces et intimidations, à constater des dégradations sur des terrains de football ou des aménagements municipaux, sans jamais pouvoir se retourner contre ceux qui dégradent volontairement ces espaces. Lorsque j'étais maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, j'ai vécu, par trois fois, des installations illicites sur mon terrain de football : elles ont eu pour conséquence une détérioration totale de cette surface, alors que la commune venait d'effectuer 30 000 euros de travaux et que les licenciés reprenaient l'entraînement. Bien sûr, puisqu'il est impossible d'attaquer un groupe, nous ne pouvons pas porter plainte, et les dégâts sont à la charge de la commune. Il faut que cela change ! Les élus doivent aussi gérer les interrogations de la population, qui fustige une justice à deux vitesses et qui considère que nos lois sont bien trop permissives. Les propriétaires privés ne comprennent pas que l'on puisse s'installer en toute impunité sur leur terrain et qu'ils doivent entamer des procédures longues. Les chefs d'entreprises sont également concernés. Des groupes s'installent par exemple sur des parkings de commerces, provoquant leur fermeture provisoire et une baisse du chiffre d'affaires. Certains chefs d'entreprise se trouvent dans l'obligation de faire appel à des services de sécurité privés. Autres professionnels lourdement importunés : les agriculteurs. Ils sont excédés, subissent des dégradations de leur outil de travail, avec toutes les nuisances que cela entraîne : pertes de récoltes, dégâts dans les champs dus aux détritus- lames de rasoir, déchets plastiques, etc. -et impact sur Je comprends ceux qui crient à l'aide et manifestent, comme récemment à Viry ou lors de la grande journée de mobilisation organisée en Haute-Savoie. J'étais, durant ces deux journées, à leurs côtés. Les gendarmes aussi sont épuisés par cette situation : face à de grands groupes, ils sont mobilisés avec des effectifs limités, pendant des périodes de plus en plus longues, alors qu'ils ont de nombreux autres dossiers à suivre. Même s'ils ont un devoir de réserve, nous pouvons aisément sentir, sur le terrain, leur exaspération. Les préfets et sous-préfets sont lassés de devoir continuellement répondre sur ce sujet aux élus locaux, à la population ou aux agriculteurs et de devoir lancer des procédures d'expulsion toujours plus nombreuses. Vous Vous l'aurez compris, madame la ministre, il y a urgence ! Urgence à légiférer sur un nouveau texte, utile et applicable, grâce auquel l'État pourra mettre des moyens à disposition. Comme je vous l'indique et comme vous l'avez déjà entendu de la part de l'ensemble des intervenants qui sont venus vous rencontrer place Beauvau, la situation est grave, très grave, et elle empire d'année en année. Nous frôlons le drame chaque semaine entre les communautés de gens du voyage et les gendarmes, élus locaux et paysans. Nous craignons que cela ne se solde par un cas mortel. La proposition de loi de mon collègue Jean-Claude Carle, dont je suis cosignataire et qui a été inspirée par le sénateur honoraire Pierre Hérisson, et celle de Loïc Hervé visant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage apportent des réponses concrètes. Je souhaite aussi remercier ma collègue Catherine Di Folco de la qualité de son rapport. Je souligne que ce texte comble un vide législatif important, en répondant aux problèmes rencontrés par les élus locaux à l'occasion des grands rassemblements et passages des gens du voyage. Veuillez conclure,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les occupations illicites sont inacceptables et les détériorations révoltantes. si toutes les émotions et la révolte que ces situations peuvent susciter sont compréhensibles, nous sommes ici, dans cette enceinte, pour voter la loi. pas pour amplifier les émotions, mais pour légiférer de manière efficace et utile. Absolument ! C'est la raison pour laquelle il nous faut commencer par dire quelques vérités.

M. Leconte a la parole. Il est absolument indispensable de faire en sorte que la loi soit respectée par l'ensemble des collectivités.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, les propositions de loi examinées aujourd'hui rappellent que l'encadrement juridique de l'accueil des gens du voyage est hautement perfectible, en raison de la sensation d'abandon ressentie par les élus, qui font face à des situations souvent critiques, généralement sources de conflits. Avec dix-sept ans d'expérience, de retours du terrain, et alors même que les élus réclament les aménagements nécessaires, la loi doit être modifiée dans l'intérêt et le respect de tous. En octobre 2016, lors de l'examen de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, le Sénat avait déjà manifesté sa volonté de rééquilibrer la loi Besson, de l'assouplir, mais sans succès face à l'Assemblée nationale, qui avait préféré le dogmatisme au pragmatisme. Alors que nous avons l'occasion de débattre à nouveau de ces enjeux un an après, j'espère que votre gouvernement, madame la ministre, se montrera, cette fois, plus à l'écoute des attentes des élus et des habitants, qui sont excédés par des comportements dépourvus de civisme,

Malgré leurs efforts, les maires sont continuellement en position d'accusés, même lorsqu'ils doivent faire face à des agissements répréhensibles, à des dégradations d'infrastructures, à des installations sauvages, voire à des comportements violents. D'une part, la question de l'évacuation est une préoccupation majeure des élus, tant sur les terrains privés que sur les aires dédiées. Face à des gens du voyage qui se déplacent de moins en moins, comme l'atteste la Cour des comptes, avec des aires permanentes d'accueil en partie détournées de leur vocation, certaines faisant même l'objet d'une appropriation par des groupes familiaux, la réponse législative actuelle est insuffisante, quel que soit le terrain. Proposer un outil juridique pour une évacuation dans les meilleurs délais, afin d'éviter que les tensions ne se cristallisent et ne deviennent encore plus difficiles à régler, tout en renforçant les sanctions, apporte un signal fort et rassurant aux élus, qui, lorsqu'ils sont face à plusieurs centaines de véhicules, n'ont pas, actuellement, de moyens d'exécution. Je pense tout particulièrement aux communes membres d'un EPCI où se situe une aire d'accueil et qui ont toujours respecté leurs engagements, ... Absolument ! ... mais qui ne peuvent plus procéder aux évacuations, car la commune voisine, appartenant pourtant au même EPCI, n'a pas rempli les siennes. Eh oui ! Pour les communes volontaires, c'est une double peine, puisque le préfet peut refuser l'utilisation de la force publique dans les communes disposant pourtant d'une aire. En l'état du droit, les gens du voyage sont définis par la loi comme les personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. À ce jour, cette définition n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni de la part des gens du voyage ni de celle des autorités publiques. C'est donc dans cet esprit que la loi doit être modifiée. D'autre part, les élus ont une marge de manoeuvre particulièrement étriquée sur le plan budgétaire. Cette compétence suscite un coût important, tant pour l'installation des emplacements légaux que pour la réparation de dégâts.

Quant à la création d'emplacements légaux, leur coût n'est pas anodin, puisque, vous l'avez rappelé, la Cour des comptes l'a estimé à près de 35 000 euros en moyenne. Même dans les communes volontaires comme Nice, où l'aire permanente, construite il y a 11 ans, est l'une des plus fréquentées de France, avec un taux de remplissage de 83 %, contre 55 % sur le reste du territoire, cette compétence représente une charge constante,

la détresse budgétaire s'accentuera dans le temps, puisque les collectivités ne peuvent plus s'appuyer, en partie, sur l'aide au logement temporaire, l'ALT, depuis qu'un décret de décembre 2014 relatif à l'aide versée aux gestionnaires d'aire d'accueil des gens du voyage a réformé ses modalités de calcul et d'attribution. Le précédent gouvernement, que j'avais interrogé sur ce point, m'avait confirmé sa volonté de moduler l'ALT en fonction du taux d'occupation des aires, alors même que, en parallèle, la Cour des comptes pointe le fait que de nombreuses aires sont peu fréquentées : entre 55 % et 60 % sont réellement occupées. Dans la mesure où des aires d'accueil sont opérationnelles, il est regrettable que les communes qui consentent à faire des efforts pour prendre à bras-le-corps ce sujet soient à nouveau pénalisées. Or forcer les maires à créer des aires d'accueil, en imposant de nouvelles contraintes financières, n'apportera pas la réponse aux blocages qui peuvent exister. Face à des frais importants, à la raréfaction des financements publics et aux risques pris à délivrer les autorisations d'installation, les communes et leurs groupements doivent avoir l'assurance que, en contrepartie de leurs efforts, elles n'en seront pas de leur poche et qu'elles auront l'appui de la force publique. La parole

qui sous-tendent les obligations faites aux collectivités territoriales de créer des lieux spécifiques. Cet accueil mérite l'attention de tous les acteurs concernés par cette problématique. problématique. Or, force est de constater que la réalité est différente : l'implication est souvent insuffisante et l'engagement financier de l'État en la matière a tendance à se réduire dangereusement. comme il est devenu effectif depuis le 1 janvier dernier, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil sont désormais une compétence des EPCI, qui deviennent les garants du respect de la loi en matière de réalisation d'aires d'accueil. S'il n'est pas incohérent que les EPCI aient désormais cette compétence, qui peut s'intégrer à celle du logement, il est en revanche très pénalisant de l'exercer sans soutien de l'État. suite de la loi Besson, pour impulser cette politique et inciter les créations d'aires, l'État avait accordé des subventions d'investissement. Aujourd'hui, ces aides ont disparu et laissent les collectivités financer intégralement cette compétence, tout en imposant des contraintes supplémentaires. La répartition de la taxe sur les résidences mobiles ne semble pas compenser les aides initialement allouées et, en tout cas dans mon département, elle est à ranger au rang des inconnues

On peut légitimement s'interroger, quand on voit le taux de fréquentation de certaines aires d'accueil. Absolument ! Sur le territoire d'une même intercommunalité, on va obliger, le cas échéant, à construire une ou plusieurs nouvelles aires, sans même se soucier de l'occupation des aires existantes. Or cela entraîne des coûts conséquents, en investissement et en fonctionnement, pour tous les partenaires. Je ne reviendrai pas sur l'investissement et n'aborderai ici que le fonctionnement. Jusqu'en 2014, l'État subventionnait le fonctionnement des aires, en octroyant une aide de 132,45 euros par place et par mois. Depuis lors, le dispositif a évolué, au détriment des collectivités territoriales, puisque, si l'enveloppe reste similaire, elle se scinde en une part fixe de 88,30 euros et une part variable de 44,15 euros versée en fonction du taux d'occupation.

La Cour des comptes constatait déjà, en 2012, que « le reste à charge pour les collectivités était significatif ». En outre, comme je l'indiquais plus haut, dans la mesure où la création est liée à un critère démographique sans lien aucun avec la présence de gens du voyage, donc avec les besoins véritables, on se retrouve devant des situations ubuesques d'aires quasiment inoccupées. Or, si cela a un coût considérable pour les collectivités, il en va de même pour l'État, qui verse une subvention fixe pour des places supplémentaires créées sans étude préalable. Des contraintes importantes, des financements gaspillés, des besoins pas satisfaits : la politique en matière d'accueil des gens du voyage a encore beaucoup à s'améliorer. Serait-ce la raison pour laquelle l'État s'en est déchargé ? Le rapport de la Cour des comptes relevait déjà, en 2012, qu'il s'agissait « d'une politique insuffisamment pilotée Outre ces questions d'infrastructures, les gestionnaires sont confrontés à des réalités, qui ne permettent pas toujours de garantir la sécurité. Le législateur a englobé, dans un terme générique, des groupes aux histoires et réalités différentes ; ce souci égalitaire, concrétisé par la terminologie, ne parvient pas, pour autant, à occulter les dissensions qui existent qui existent entre communautés. Leur cohabitation est souvent difficile, source de tensions, en raison de modes de vie et de pensée bien différents. Actuellement, l'arrivée de populations nombreuses d'Europe de l'Est, notamment croates, génère pour les gestionnaires d'aires d'accueil de grandes difficultés. Celles-ci sont accrues, dans certaines communes, que les forces de police nationale ou municipale refusent de rentrer sur les aires d'accueil, arguant de leur caractère privé, alors même que les maires ont conservé le pouvoir de police et que l'État est censé intervenir partout. Ici, comme dans certains

Louis Masson, sur l'article. Madame la présidente, je voudrais souligner les problèmes que me pose ce texte, notamment son article 1, en ce qui concerne les rapports entre les communes et les intercommunalités. des raisons d'équité, il revient avant tout aux communes de plus de 5 000 habitants de créer des aires d'accueil. Or, avec le transfert obligatoire, notamment dans le cas des communautés d'agglomération, de la compétence

Avec un tel système- donner à l'intercommunalité la possibilité de choisir une petite commune d'une aire de nomades, qui normalement devrait se situer dans une commune de plus de 5 000 habitants -, on aboutit à des situations profondément injustes, car ce sont toujours

j'ai pu remarquer la grande sagesse dont celui-ci a toujours fait preuve, considérant que, dans cette affaire, il fallait que les communes et les intercommunalités respectent leurs droits et leurs devoirs, de même qu'il fallait que les gens du voyage respectent leurs droits et leurs devoirs.

en matière de terrains d'accueil et de terrains de grand passage. Par ailleurs, il est clair qu'il faut renforcer les moyens des maires et des présidents d'intercommunalité pour faire appliquer la loi lorsque ces terrains existent. Nous

un grand nombre d'articles inspirés par Dominique Raimbourg, qui s'inscrit exactement dans la même philosophie que Louis Besson. Tout le monde sait que cette loi a été adoptée après de longs débats

Nous, nous ne l'avons pas adoptée ! Madame Gatel, cette loi a été adoptée par le Parlement, en vertu de la Constitution de la République française. Elle est donc parfaitement adoptée, même si vous ne l'avez pas votée ! Nous devons respecter la loi, même si nous ne l'avons pas votée. Cette loi

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à l'approche de votre déplacement en Guadeloupe, le 4 novembre les questions de l'emploi et des déchets, tout comme celles de l'alimentation en eau potable et des transports, constituent les principales préoccupations des Guadeloupéens. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la problématique du financement des investissements dans l'eau potable en Guadeloupe, ce que l'on appelle dans ma région « le scandale de l'eau Les coupures d'eau sont désormais quotidiennes en Guadeloupe. Karukéra, l'île aux belles eaux, est devenue l'île sans eau ! Cette question est préoccupante dans un pays où le précieux liquide ne semble pourtant pas manquer. En effet, si nous ne souffrons pas d'une production insuffisante, l'état désastreux des réseaux et des installations connexes nous indique l'ampleur de la catastrophe. De façon systématique, des coupures d'eau ont lieu dans les communes. Elles sont appelées « tours d'eau ». Ces coupures touchent et handicapent la quasi-totalité de la population. Le rendement du réseau est, en moyenne, à moins de 50 %. Nos réseaux demeurent archaïques, datant pour la plupart de plus de cinquante ans. De nombreuses études sur la question du volume des investissements à réaliser ont affaires régionales, le SGAR, de 2016, s'accordent à admettre qu'il nous faudra, sur les dix années à venir, mobiliser plus de 900 millions d'euros afin de mettre aux normes nos installations. Monsieur le Premier ministre, vous le comprendrez, cette situation doit changer ! La question de l'eau est un enjeu à la fois économique, environnemental et sanitaire. Comment admettre, en 2017, dans une île tournée vers un tourisme de qualité, gage de son développement, nous puissions assister à de tels « tours d'eau » et que certains foyers se trouvent privés d'eau plus de quatre jours dans la semaine ? Malgré les efforts financiers des collectivités locales, nous sommes très loin des montants nécessaires à la résolution de ce problème. Ma question sera donc la suivante : pouvez-vous nous indiquer quelles sont les différentes mesures d'aide que prendra le Gouvernement sur cette question, dans le cadre d'une véritable solidarité nationale ? Rappelons que, dans son programme présidentiel, le candidat Macron, devenu Président de la République, indiquait qu'un milliard d'euros seraient consacrés à la Guadeloupe sur les cinq prochaines années, afin de résoudre les problèmes d'eau et d'assainissement. La parole

Il n'est pas tolérable, ni pour vous ni pour nous, qu'une partie de la population française subisse des coupures d'eau quotidiennes. Par conséquent, depuis plusieurs années, l'État et ses opérateurs apportent d'ores et déjà un appui technique et financier important aux collectivités locales, qui sont, comme vous le savez, compétentes en matière d'alimentation en eau potable, afin de les aider à améliorer la situation. est vrai que la géographie de l'île et ses conditions climatiques rendent parfois difficile l'accès à la ressource en eau, qui ne manque pas, comme vous l'avez évoqué, d'où la nécessité d'infrastructures pour l'acheminer là où il y en a besoin. Des investissements sont ainsi en cours pour la réalisation d'opérations prioritaires, d'améliorer les infrastructures. Des financements importants- plusieurs dizaines de millions d'euros -sont par ailleurs mobilisables jusqu'en 2020 les fonds européens, les crédits d'État, l'Office de l'eau et le conseil régional. Toutefois, l'argent n'est pas le facteur limitant. C'est sa mobilisation, qui doit permettre l'émergence de projets opérationnels opérationnels et finalisés, qui est difficile. Partant du diagnostic qui a été dressé par un rapport interministériel, l'État a donc lancé un Plan national d'action pour les services d'eau et d'assainissement en Guadeloupe et

Mon secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, qui travaille avec moi sur ce sujet, ira sur place en fin de semaine à l'occasion du déplacement du Premier ministre. Ce sera l'occasion de tirer les enseignements du passé, afin de poursuivre le travail mené en soutien aux collectivités

et Social Européen. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre et concerne la gouvernance des aéroports régionaux, plus particulièrement celui de Toulouse-Blagnac. Le décret d'avril 2015 a permis au consortium chinois Casil Europe d'entrer au conseil d'administration à hauteur de 49,99 % du capital. Les actionnaires publics locaux- conseil départemental, région Occitanie, Toulouse Métropole, chambre de commerce et d'industrie -s'étaient alors inquiétés de l'évolution de la gouvernance de cet outil de développement essentiel pour le territoire, infrastructure de transport hautement stratégique, y compris pour Airbus qui en est un utilisateur privilégié. Aujourd'hui, c'est l'avenir des dernières parts de l'État qui cristallise les appréhensions, puisque le décret dispose qu'une option de vente pourrait être exercée, dès 2018. Ce sujet d'inquiétude s'est trouvé renforcé par les prises de position des actionnaires privés en conseil d'administration. Si 12,8 millions d'euros ont été redistribués aux actionnaires au titre des bénéfices des exercices 2015 et 2016, ce sont 15 millions d'euros de plus qui leur ont été versés en 2017 sur les réserves financières de l'aéroport. Il me semble que ces dernières n'ont pas vocation à rémunérer un investisseur privé. Compte tenu de ces éléments et des craintes unanimes des acteurs publics locaux et des industriels, pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, nous assurer que les dernières parts détenues par l'État ne feront pas l'objet d'une vente au consortium privé déjà présent, garantissant ainsi une minorité de blocage de 50,01 % pour les acteurs publics- à moins que tout cela ne soit déjà inscrit dans le pacte des actionnaires qui n'a, hélas, jamais été rendu public ? La parole

L'État a gardé 10,01 % de ses parts et ne peut pas les vendre avant avril 2018. Je voudrais juste vous rassurer sur un certain nombre de points. Tout d'abord, s'il y a eu versement de dividendes, y a eu versement de dividendes, c'est parce que l'aéroport se porte bien. Si l'État actionnaire a accepté ce versement, c'est tout simplement parce que les résultats sont bons et qu'il y a des investissements- 160 millions d'euros d'investissements prévus pour l'aéroport de Toulouse, c'est une excellente nouvelle

s'agissant des parts de l'État- 10,01 % -, je peux vous assurer qu'aucune décision ne sera prise sans concertation étroite avec les élus locaux, avec la région, avec le département, avec vous-même, madame la sénatrice, ... Merci ! ... avec les communautés de communes, la ville de Toulouse et, évidemment, avec les entreprises représentées dans le cadre de la chambre de commerce. Nous sommes rassurés, alors ! Nous connaissons parfaitement la sensibilité du sujet. L'aéroport de Toulouse est un magnifique projet industriel, il se porte bien, il a des investissements et il est lié à l'avenir d'Airbus, qui nous tient aussi extrêmement à coeur. Soyez rassurée, aucune décision ne sera prise sans une concertation étroite avec les élus locaux et sans la certitude qu'elle va dans le sens de l'intérêt général.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues sénatrices et sénateurs, en novembre 2015, l'Agence européenne de sécurité des aliments a rendu un avis sur le glyphosate et considéré que « son potentiel cancérigène était improbable Le 13 avril 2016, le Parlement européen a demandé la divulgation sans délai des données scientifiques de cette expertise. Cette demande de transparence et de contrôle démocratique, qui touche au principe de précaution, est restée lettre morte. Le 5 octobre dernier, notre collègue Sabine Thillaye, présidente de la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, s'est interrogée sur « l'indépendance et l'objectivité des agences européennes chargées d'évaluer la dangerosité des substances mises sur le marché » et a saisi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur ce sujet. Dans une résolution du 24 octobre dernier, le Parlement européen a rappelé une nouvelle fois que « l'évaluation scientifique des pesticides [doit s'appuyer] uniquement sur des études publiées indépendantes, ayant fait l'objet d'un examen par des pairs et commandées par les autorités publiques compétentes Le 10 octobre dernier, le commissaire européen Phil Hogan a déclaré à propos du glyphosate : « Notre science montre qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine ». Mais de quelle science s'agit-il ? Celle des entreprises mondiales, nouvelle inquisition du XXI siècle, qui n'acceptent que les preuves scientifiques conformes à leurs intérêts et excommunient les chercheurs qui les contestent La Commission européenne discutera le 9 novembre prochain du renouvellement de la licence du glyphosate. À tout le moins, il nous semblerait illégitime qu'elle se prononçât à partir d'un avis scientifique suspecté d'insincérité. Nous vous demandons, monsieur le ministre, de défendre devant cette instance les dernières résolutions du Parlement européen, notamment l'élimination progressive et définitive du glyphosate avant 2022. La parole est à M. le ministre d'État,

tellement que l'application du principe de précaution me semble tout à fait d'actualité. La semaine dernière, les États membres ont effectivement refusé de réautoriser pour dix ans le glyphosate.

une agence de l'Organisation mondiale de la santé, qui, elle, ne s'est jamais trompée dans son diagnostic et a bien dit que le glyphosate était un « cancérogène probable ». D'autres informations convergent vers nous et je ne pense pas que nous puissions prendre de risque avec la santé. N'attendons pas la démonstration du pire pour mettre effectivement en oeuvre le principe de précaution. La position du Gouvernement

qui, à juste titre, se sentent parfois prisonniers du glyphosate. Et de l'opinion ! J'en suis convaincu, nous allons prendre le temps de faire émerger des alternatives. Certaines existent déjà, d'autres sont « dans les tuyaux », notamment La priorité absolue, aujourd'hui, est bien de valoriser ces initiatives, de les identifier et de les partager

raison du choix désormais possible entre la semaine de 4 jours et celle de 4 jours et demi. Très sollicités par les enseignants et les parents d'élèves, les maires sont confrontés à ce choix, avec un élément important à considérer dans la décision qu'ils auront à prendre : le coût à assumer pour la collectivité. Ce coût suscite des interrogations, voire de l'inquiétude, pour les élus locaux et, plus généralement, pour tous les acteurs concernés par cette réforme. Or pour les territoires qui ont parfaitement joué le jeu de cette nouvelle organisation, et qui s'en déclarent très satisfaits, la poursuite des nouvelles activités périscolaires doit pouvoir s'effectuer dans les meilleures conditions d'accueil, avec une offre de qualité, et ce dans l'intérêt supérieur des enfants. Cela nécessite de la visibilité quant au type d'accompagnement financier. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je voudrais savoir quel sera, pour l'année scolaire 2018-2019, l'accompagnement financier pour les communes qui maintiennent la semaine de 4 jours et demi et les activités périscolaires qui l'accompagnent.

après, il est vrai, beaucoup de discussions, pour ne pas dire des incitations très fortes. Monsieur le ministre, envisagez-vous de défendre auprès de la CAF le principe de la poursuite de ces aides indispensables ?

effet une question importante de cette année scolaire, mais aussi de l'année suivante, puisque c'est en ce moment que les maires, avec les communautés éducatives, prennent ces décisions. Je vous remercie de cette question qui est tournée vers l'avenir, donc vers la qualité de ce qui va se passer pour l'organisation scolaire.

Il est programmé, en loi de finances pour 2018, pour 237 millions d'euros, avec un calcul qui est le même que précédemment, c'est-à-dire 50 euros par élève et 90 euros en zone d'éducation prioritaire. C'est donc un effort dans la continuité qui est réalisé par l'État. Cela vous montre bien, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'incitation à passer à 4 jours, mais tout simplement, je le répète, une continuité de la parole en la matière. Dans les temps qui viennent, nous serons concentrés sur l'enjeu de la qualité de ce qui se passe en matière périscolaire. Les moyens sont là et, vous l'avez dit, il est important aussi d'être attentif aussi à la question des moyens donnés par les caisses d'allocations familiales. Nous menons un dialogue avec la caisse nationale, et j'observe de la bonne volonté. Je suis donc assez optimiste sur le fait que nous aurons au moins les mêmes moyens l'an prochain sur cette question. Toutefois, nous allons progresser sur deux points au moins. Le premier, c'est la simplification des procédures. Tout le monde la souhaite, et nous sommes en train d'y travailler. Le second, c'est peut-être l'amplification de l'aide, avec une veille sur la qualité de ce qui se passe.

qui se tient aujourd'hui, inquiet, devant vous. En juin dernier, vous avez laissé la liberté d'organiser la semaine scolaire école par école. Dès septembre, 44 % des communes ont décidé de quitter le dispositif des rythmes scolaires. Aujourd'hui, des académies demandent aux maires de se prononcer dès le 15 décembre pour la rentrée prochaine. Faire, défaire, il faut savoir tenir le rythme Selon Jules Ferry- pour ne citer que lui, qui fut aussi président du Sénat -l'école solidarise les territoires. Or il est clair que, aujourd'hui, le sillon des inégalités territoriales se creuse.

Modifier les rythmes scolaires, vous le savez, c'est changer la vie non seulement des enfants, mais aussi des enseignants et des employés municipaux, ainsi que l'organisation de la vie familiale et professionnelle.

valeur, et d'autres qui se trouvaient dans une situation totalement désespérée. C'est pourquoi plus de 40 % d'entre elles ont saisi l'occasion de ce décret pour passer à 4 jours. Personne ne les a obligées, et, comme je l'ai dit précédemment, le fonds n'est que pour celles qui restent à 4 jours et demi. Même avec cette incitation, les communes ont donc malgré tout choisi 4 jours. C'est une philosophie. Jules Ferry, que vous avez cité, disait que le principe d'autorité est ce qui est à l'opposé de l'humanisme et de la République. Justement, nous ne sommes pas dans le principe d'autorité, ni dans l'argument d'autorité ; nous sommes dans l'argument de liberté. Il appartient aux communautés éducatives de choisir ce qui leur va.

et le mercredi. Certaines communes s'en sortiront bien à 4 jours, d'autres à 4 jours et demi. C'est cela le pragmatisme, c'est cela la liberté

à grand renfort de publicité, un choc sur l'offre de logements. Or les mesures que vous venez de faire voter à l'Assemblée nationale dans la loi de finances vont provoquer un contre-choc sur cette offre. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en décidant, notamment,

vous allez mettre à l'écart 70 % du territoire national, représentant toutes les villes moyennes et toute la ruralité de notre belle France. C'est une décision tout à fait funeste.

Le PTZ, tel que nous l'avons fléché aujourd'hui, comprend d'abord le maintien à 40 % sur l'ancien sur toutes les zones B2 et C, ce qui est significatif, car c'est là où il y a le plus besoin d'accession dans le bâti ancien. Sur le neuf, nous l'avons prévu sur 2 ans, à 20 % effectivement, mais je crois qu'il s'agit d'un équilibre tout à fait opportun, qui ne va pas susciter les conséquences que vous nous avez indiquées.

et vers les rénovations des passoires énergétiques. J'ajoute, et je pense que vous y serez tout à fait sensible, que nous présenterons dans les prochains mois le plan « villes moyennes », sur lequel Action Logement interviendra de manière assez importante, une fois que la convention sera signée. Ces trois éléments

en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les acteurs calédoniens sont d'ailleurs à Paris cette semaine, et je souhaite une issue positive à la réunion du Comité des signataires de l'accord de Nouméa, ce jeudi. Nous le savons, madame la ministre, vous mesurez à quel point la situation est explosive, pour ne pas dire plus, à Mayotte. Plus que jamais, l'outre-mer est un sujet d'attention positive, mais aussi de préoccupation pour notre pays. Dans ces contextes localement compliqués, dans une période de disette budgétaire et de volonté de refondation de nos politiques publiques à l'échelle nationale, le Président de la République a défini, à l'occasion de son déplacement en

cela ne définit pas positivement ce qu'est la vision de l'outre-mer aux yeux du Gouvernement. Madame la ministre, alors que les assises des outre-mer s'annoncent, pouvez-vous nous éclairer sur cette question ? La parole est à Mme la ministre des outre-mer.

un dernier étage, constitué de 35 mesures, qui avaient été pensées unilatéralement par les membres du collectif, et sur lesquelles il faut travailler, projet par projet, mais avec les collectivités territoriales. Tel est le nouveau message du Président de la République. Il nous faut coconstruire sur les territoires des réponses à leurs difficultés,

et Social Européen. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adressait à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Plusieurs centaines de plaintes viennent d'être déposées par les utilisateurs du Lévothyrox dans le cadre de l'enquête sur la nouvelle formule. Une perquisition a été menée au siège de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Cette affaire prend donc aujourd'hui une tournure judiciaire. Nous en connaissons les contours depuis sa forte médiatisation l'été dernier. Je les rappelle : plus de trois millions de Français, dont 2,5 millions de femmes, sous prescription ; un changement de formule en mars 2017 par le laboratoire Merck plusieurs milliers de patients gênés, voire handicapés, parfois gravement, par la nouvelle formule. Face à ces problèmes et à la demande pressante des patients pour un retour à l'ancienne formule, la ministre des solidarités et de la santé a récemment annoncé que cinq nouveaux médicaments seraient disponibles. C'est une bonne nouvelle, mais que de temps perdu pour les patients, qui ont donné l'alerte sur les inconvénients de la nouvelle formule alors que ce problème aurait dû, me semble-t-il, surgir des instances de pharmacovigilance. Monsieur le secrétaire d'État, à ce stade, sans vouloir préjuger des résultats de l'enquête, que savons-nous des responsabilités des acteurs impliqués dans la chaîne de surveillance des produits de santé ? La parole

Vous l'avez indiqué, c'est au mois de mars dernier que le principe actif a été considéré comme devant faire l'objet d'un changement et que le nouveau produit a été proposé à la vente. Près de 15 000 personnes ont été identifiées comme ayant présenté des souffrances graves, lesquelles se sont exprimées à partir du début du mois de juillet, jusqu'au mois d'août dernier. La ministre a très vite diligenté une enquête, une inspection, un contrôle, compte tenu des premiers symptômes, tels qu'ils étaient apparus. Cette enquête a permis de montrer qu'il y avait effectivement des dysfonctionnements

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a suscité beaucoup d'espoir chez tous ceux qui déplorent que l'université française n'arrive plus à se hisser au même niveau que ses homologues à l'étranger. Le taux d'échec des étudiants grandissant- ils sont moins d'un tiers à réussir leur licence en trois ans -, le Président de la République n'a-t-il pas déclaré : « Il faut arrêter de croire que l'université est la solution pour tout le monde » Les Français, à plus de 66 %, sont conscients également de l'absurdité d'un système éducatif qui tourne le dos au mérite. Ils sont prêts à entendre la vérité. Aussi, pourquoi éviter les mots « prérequis » et « sélection » sont prêts à entendre, monsieur le Premier ministre, que l'université n'est pas la solution pour tout le monde, car la pire des sélections est la sélection sociale. C'est vrai ! Votre idée, c'est vous qui le dites, n'est pas de dire « oui ou non », mais de dire « oui ou oui si » et de donner le dernier mot aux étudiants. Bel exercice sémantique qui fleure bon la prudence, peut-être même le compromis ... Ne pensez-vous pas, monsieur le Premier ministre, que le mérite, que je qualifie de républicain, doit être le critère déterminant pour orienter les étudiants et assurer l'égalité entre les citoyens ? Ne pensez-vous pas qu'en euphémisant votre projet initial et en cédant devant ceux dont l'idéologie a mis à mal notre système éducatif depuis de trop longues années, ... C'est vous qui l'avez mis à mal ! ... vous risquez de faire rater à la France, à l'université et à ses étudiants une belle occasion de réforme

en examinant peut-être moins qu'il ne le fallait la réalité de l'enseignement supérieur. La réalité de l'enseignement supérieur, quelle est-elle aujourd'hui ? Elle est une sélection massive par l'échec ; elle est une sélection injuste par le tirage au sort. disant cela, je décris une réalité qui n'est pas satisfaisante et qui même, à certains égards- pardon d'employer ce terme -, n'est pas glorieuse. Elle n'est pas glorieuse collectivement, s'agissant d'un dispositif qui est pourtant essentiel à l'avenir de notre pays, à la formation de sa jeunesse, au relèvement du défi de l'intelligence collective, au relèvement du défi individuel de l'épanouissement par l'intelligence. Au total, nous obtenons des résultats qui ne sont pas glorieux. Certes, il y a encore de remarquables résultats à l'université et dans l'ensemble de l'enseignement supérieur français, bien entendu, mais 60

J'ai voulu, avec la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et avec le ministre de l'éducation nationale, concevoir un système qui permettrait d'apporter des réponses crédibles à ces dysfonctionnements, en faisant le pari de l'orientation et de de l'association des enseignants du second degré et des enseignants du supérieur à la définition de ce qui est nécessaire pour que l'étudiant réussisse. Nous avons fait le pari de la réussite pour les étudiants ! Cela passe par une meilleure orientation lors du second cycle cycle et par une meilleure information sur la réalité des filières, sur leurs succès et sur ce qui est attendu d'un étudiant. Ainsi celui-ci aura-t-il les meilleures chances de réussir dans la filière qu'il aura choisie.

de l'accompagnement, des moyens supplémentaires aussi, à savoir un milliard d'euros si l'on additionne les fonds au titre du grand plan d'investissement et les crédits budgétaires mis à disposition des établissements d'enseignement supérieur dans les cinq années qui viennent.

que leur parcours s'effectue dans de meilleures conditions. C'est le sens de la suppression de la cotisation de sécurité sociale étudiante et du rattachement de l'ensemble des étudiants au régime général de la sécurité sociale, pour rendre un meilleur service,

de l'intérieur. Monsieur le ministre, l'État islamique a perdu une bataille. De ses fiefs de Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak, il ne reste plus que des villes ravagées et des populations anéanties. Mais les terroristes n'ont pas dit leur dernier mot. Le pire est sans doute à venir : partis en Syrie pour combattre aux côtés de Daesh, un couple et ses trois enfants souhaitent être rapatriés en France après avoir été capturés par les Kurdes du PKK à Raqqa. dizaines de combattants seraient déjà revenus sur notre territoire, peut-être prêts à commettre l'irréparable, une horreur que nous ne voulons pourtant plus revoir. Combien sont-ils, monsieur le ministre ? Comment sont-ils revenus ? Sont-ils bien surveillés par nos services de renseignement ? Comptez-vous mettre en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour traduire les djihadistes français en justice et les mettre hors d'état de nuire ? Que comptez-vous faire de ces enfants et adolescents, partis avec leur famille ou nés au Moyen-Orient, qui ont connu l'horreur ou parfois commis les pires atrocités ? Souvenons-nous que près de 240 de nos compatriotes ont déjà perdu la vie dans les attentats commis sur notre propre sol. Vous devez aux Français la protection à laquelle ils aspirent légitimement. Vous devez aux Français une action résolue, impitoyable et sans merci. L'avenir de notre civilisation est en jeu. N'attendons pas le pire pour agir ! Je vous remercie, monsieur le ministre d'État, de nous éclairer sur les actions que le Gouvernement entend mener pour lutter avec la plus grande efficacité face à cette nouvelle étape de notre guerre contre le terrorisme. La parole

la sénatrice Darcos, le combat contre le terrorisme est notre priorité. Il est la priorité du Gouvernement, mais il est notre priorité commune. Aujourd'hui, vient d'entrer en vigueur la loi que nous avons adoptée ensemble pour combattre le terrorisme. Je veux remercier les sénateurs

-, 58 mineurs. La plupart des majeurs sont sous main de justice. Très exactement, 120 hommes, sur les 178, ont été écroués et sont aujourd'hui en prison. Les autres sont suivis par la DGSI,

Vous avez raison, il s'agit d'un combat global, d'un combat de civilisation. Nous, nous sommes pour la liberté, la liberté des femmes et des hommes dans le monde ; nous ne sommes pas pour le retour à des théories barbares et primitives.

Les Landes- comme d'autres départements du sud-ouest de la France -ont été durement impactées par deux phases consécutives de grippe aviaire. Des centaines de producteurs de palmipèdes et de volailles ont souffert et souffrent encore face à cette crise d'ampleur inédite. La filière tout entière, de l'amont à l'aval, est concernée. Cela représente, sur le territoire landais, plus de 5 000 emplois. Si un certain nombre d'aides ont été apportées sous le gouvernement précédent par l'État et par l'Europe, un problème majeur subsiste la date de fin du vide sanitaire a été arrêtée au 29 mai 2017. Les pertes d'exploitation sont donc couvertes jusqu'à cette date ... Mais cette date ne peut être que théorique. En effet, toute la chaîne ayant été touchée, y compris les fournisseurs de reproducteurs et de canetons, les élevages ne reviennent en fonctionnement que petit à petit, sur plusieurs semaines. Il faut donc prévoir une couverture des pertes d'exploitation qui va au-delà du 29 mai. Une mobilisation de la filière mais aussi de plus de 200 élus a eu lieu le samedi 14 octobre. Parce que nous devons soutenir des familles qui vivent aujourd'hui des situations très compliquées, et parce que la filière agroalimentaire est une des principales richesses de notre département. À l'occasion des fêtes de fin d'année, j'espère que nombre d'entre vous dégusteront du foie gras, mets d'excellence particulièrement ancré dans notre tradition culinaire et gastronomique. N'oublions simplement pas que pour maintenir la production de ce que Henri Emmanuelli appelait « le pétrole des Landes et par là même les 5 000 emplois induits, il faut soutenir les producteurs et la filière dans son ensemble. C'est pourquoi, monsieur le ministre, si l'ouverture du dispositif d'indemnisation de l'aval de la filière palmipèdes vient d'être annoncée pour 2016, nous attendons une réponse claire sur l'indemnisation des producteurs au-delà du 29 mai 2017. La parole

Concernant la crise de 2007 H5N8, les paiements pour indemniser les abattages préventifs subis dans les élevages sont pratiquement achevés aujourd'hui à hauteur de 13 millions d'euros. le dispositif qui permet le versement d'une avance de 50 % sur les pertes de non-production dans les zones réglementées a débuté à la mi-juin et est en cours de règlement sur 95 % des dossiers. Comme je l'avais annoncé le 23 juin dernier, une seconde avance de 20 % a été octroyée. Les paiements ont démarré depuis la deuxième quinzaine d'octobre. S'agissant du maillon « sélection et accouvage », un nouveau dispositif qui permet la prise en charge des pertes par les accouveurs est déployé depuis le début du mois d'août. Les paiements devraient intervenir, pour eux, à partir du mois de novembre.

de tenter une médiation pour savoir si nous sommes en mesure d'ouvrir une indemnisation sur ces pertes indirectes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de retour particulier, mais nous essayons d'avancer et de trouver des solutions pour faire en sorte que ces pertes indirectes puissent être

Ainsi, la France a retrouvé son statut « indemne » sur l'influenza aviaire, ce qui a permis au Japon de rouvrir son marché aux produits de volailles et au foie gras, et je m'en réjouis, bien évidemment, pour l'ensemble de la filière du Sud-Ouest. La

j'ai pu constater qu'une question était prioritairement évoquée par les présidents d'intercommunalité. Elle concerne le Fonds national de péréquation des ressources

contributrices en majorité au profit des intercommunalités urbaines, c'est surtout l'application du coefficient qui varie de 1 à 2- vous avez bien entendu, mes chers collègues, de 1 à 2 ! -en fonction du nombre d'habitants, au motif que, plus il y a d'habitants, plus il y a de charges.

Madame la ministre, si on ne veut pas exacerber les clivages entre milieu rural et milieu urbain, il faut revenir sur ce coefficient de 1 à 2, qui est injuste et injustifié. Ma question est donc simple : allez-vous prendre des mesures pour revenir à l'équité ?

pour les calculs faits sur la base de ressources consolidées d'effet anti-péréquateur, nous avons aménagé des mécanismes qui permettent de traiter la question des communes riches dans un ensemble intercommunal pauvre et vice versa.

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, je vous remercie. Je rappelle que les prochaines questions d'actualité au Gouvernement

de la discussion de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage, présentée par M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues, en examen conjoint avec la proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé, présentée par M. Loïc Hervé et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion du texte de la

En outre, la mesure proposée qui consisterait à conditionner la réalisation des aires et des terrains familiaux et de grands passages sur la base d'un nouvel indicateur correspondant à un taux d'occupation minimal de l'offre existante introduirait une nouvelle norme inappropriée et inopérante.

Pour mémoire, les communautés de communes ne comportant que des communes de moins de 5 000 habitants représentent près de 45 % des communautés sur le plan national. On ne saurait donc les exonérer de leur compétence en matière d'accueil des gens du voyage, au risque d'alléger considérablement le volume global des obligations qui leur incombent au titre de la loi de 2000. Il est par ailleurs proposé de fixer comme critère supplémentaire de détermination celui d'un taux d'occupation des aménagements existant dans le même secteur géographique. Même si l'on comprend l'intention qui sous-tend cette disposition, une telle mesure reviendrait à complexifier le dispositif actuel de manière inutile dès lors que le schéma départemental, fait en concertation entre l'État et le conseil départemental, s'appuie nécessairement sur une évaluation réelle des besoins. Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer les alinéas 3 à 6 du présent article.

le principe de portée générale inscrit dans la loi du 5 juillet 2000, selon lequel « les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage ». Ce principe est reconnu de longue date par la République et l'aménagement des aires et terrains d'accueil prévus par les schémas départementaux n'est que l'une de ses modalités d'application. Les communes non inscrites au schéma et dépourvues d'aires d'accueil sont tenues, elles aussi, de « participer à l'accueil des gens du voyage » en les laissant stationner quelques heures sur leur territoire- sauf si elles appartiennent à un EPCI qui a rempli les obligations mises à sa charge Substituer à ce principe général la disposition selon laquelle les « établissements publics de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs communes de plus de 5 000 habitants participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage » constituerait donc un recul pour les droits de ces personnes. personnes. On peut s'étonner aussi que votre groupe, monsieur Collombat, supprime la disposition selon laquelle le préfet peut signer seul le schéma, si le président du conseil départemental refuse de le faire. En effet, cette disposition est indispensable pour empêcher des blocages. élément, l'amendement fait l'impasse sur les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage, alors qu'ils figurent au schéma. Ces terrains et ces aires sont évidemment indispensables.

et 28, qui sont contraires à la position de la commission. En premier lieu, ils visent à supprimer la disposition selon laquelle le schéma départemental ne peut prévoir, à titre obligatoire, la réalisation d'aires ou de terrains d'accueil dans les petites communautés de communes rurales ne comportant aucune commune de plus de 5 000 habitants. est conforme à l'intention du législateur de 2000, puisqu'il n'envisageait la création d'aires d'accueil que dans les « agglomérations ». Elle met le droit en accord avec la pratique, puisque les schémas départementaux que l'on a pu consulter n'imposent pas d'obligations à de telles communautés de communes. Il arrive que le schéma prévoie, à titre facultatif, la réalisation d'aires ou de terrains d'accueil dans les EPCI ne comportant aucune commune de plus de 5 000 habitants, la commission a eu soin de conserver cette simple faculté. Ce n'est pas une interdiction stricte, il subsiste la faculté de le faire. En second lieu, les amendements visent à supprimer la disposition introduite en commission sur l'initiative de Mme Gatel, selon laquelle le schéma départemental ne peut prévoir la création de nouvelles aires ou de nouveaux terrains si le taux d'occupation des aires et terrains existant dans le même secteur géographique d'implantation est inférieur à un seuil défini par décret. On voit mal pourquoi les communes et leurs groupements créeraient de nouvelles aires ou de nouveaux terrains si ceux qui existent aux alentours restent à moitié vides

Je ne peux pas laisser dire cela ! Quelle est la situation actuelle ? La loi Besson prévoit que ne sont assujetties à l'obligation de participer au schéma que les communes de plus de 5 000 habitants.

les collectivités territoriales en prévoyant de comptabiliser dans le taux de logements locatifs sociaux les emplacements des aires permanentes d'accueil des gens du voyage. En effet, ces aires permanentes d'accueil entrent pleinement dans le champ des hébergements sociaux puisque ce sont des lieux de séjour qui peuvent accueillir des personnes en situation de précarité et que celles-ci peuvent rester sur ces lieux plusieurs mois, voire plusieurs années. De plus, ces aires représentent un coût non négligeable pour les collectivités locales qui en ont la charge. Ce sont des équipements pérennes et qui sont à la fois construits et gérés par les collectivités locales, avec un accès aux commodités. Enfin, je rappelle que les dépenses, notamment foncières, faites par une commune pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage peuvent déjà être déduites au titre des pénalités de la loi

puisque ces aires, comme les logements sociaux, sont destinées à des personnes qui sont souvent en situation de précarité, que leur création, leur aménagement, leur entretien et leur gestion coûtent cher aux communes et EPCI et que les dépenses exposées à ce titre par les communes et leurs groupements sont déjà déductibles du prélèvement sur les ressources fiscales des communes qui n'ont pas atteint le taux de logements sociaux prévu par la loi SRU.

et à l'habitat des gens du voyage. Il a toujours été considéré que les aires d'accueil des gens du voyage ne sauraient être assimilées à des logements pérennes destinés à des ménages modestes et dont la production nécessaire constitue l'essence même des dispositions de l'article 55 de la loi SRU. Elles ne sauraient donc être décomptées au titre de cette loi, et ce d'autant moins que, en l'absence de bail ou d'occupation de type locatif, aucun mécanisme ne vient garantir l'occupation effective de ces aires à des fins sociales par des personnes sous plafond de ressources, ce qui rendrait impossible une comptabilisation permettant de vérifier la satisfaction des objectifs SRU.

que doivent remplir les communes. Je ne comprends pas la logique qui préside au refus du Gouvernement de les considérer comme des logements sociaux de fait. Tous les

À mes yeux, ces aires entrent pleinement dans le champ des hébergements sociaux.

l'amendement n° 22. Il s'agit d'un amendement de suppression. Nous considérons que l'article 2 est un encouragement à l'immobilisme. Il vide de sa substance le pouvoir de substitution du préfet aux communes et aux EPCI qui ne respectent pas le schéma départemental d'accueil des gens du voyage en réduisant son champ d'application et, surtout, en supprimant le dispositif de consignation de fonds auquel il est adossé.

relative à l'égalité à la citoyenneté. Il constitue une amélioration du dispositif d'accueil des gens du voyage dans la mesure où il permet au représentant de l'État dans le département de prendre des mesures efficaces et pratiques lorsque les obligations prévues par le schéma départemental n'ont pas été accomplies par les communes ou les EPCI. Il ne s'agit pas d'une mesure coercitive, il s'agit d'une disposition incitative, de bonne application de la loi, que le préfet peut utiliser avant, éventuellement, de mettre en oeuvre le mécanisme de substitution prévu à l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 En outre, l'introduction récente du mécanisme de consignation ne laisse aucun recul sur l'efficacité de sa mise en oeuvre. Il est donc particulièrement inopportun, à notre avis, de le supprimer.

de mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Contrairement à ce qu'a dit M. Fichet, la commission n'a pas remis en cause la possibilité pour le préfet de se substituer à une commune ou un EPCI défaillant, que les précisions apportées par la loi « égalité et citoyenneté » sur les modalités d'application de cette procédure de substitution. Nous n'y touchons pas. La commission a seulement estimé que la procédure de consignation de fonds était inutilement attentatoire attentatoire à la libre administration des collectivités territoriales. Si le préfet se substitue à une commune ou à un EPCI, les dépenses qu'il engage pour réaliser des aires ou des terrains d'accueil constituent des dépenses obligatoires pour cette commune ou cet EPCI. Il suffit donc à l'État de faire l'avance des fonds.

Il vise donc à faire obligation aux responsables du convoi d'avertir les autorités locales vingt-quatre heures avant l'arrivée sur les lieux. Cette mesure permettra d'anticiper au mieux l'accueil des personnes dites « gens du voyage » et d'organiser leur arrivée et leur stationnement.

il devrait être notifié au maire au moins vingt-quatre heures à l'avance. Le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur la faculté d'apporter des restrictions aux libertés constitutionnellement garanties, telles que la liberté d'aller et venir, afin de les concilier avec d'autres objectifs de valeur constitutionnelle, tels que le maintien de l'ordre public. Ces restrictions peuvent notamment consister en un régime d'autorisation ou de déclaration préalable. Toutefois, on peut s'interroger sur la proportionnalité de la mesure proposée, d'autant qu'aucun seuil n'est fixé : n'importe quel groupe de caravanes, fût-ce de deux unités, devrait, avant de stationner sur le territoire d'une commune, en informer le maire au moins vingt-quatre heures à l'avance. Il n'est d'ailleurs pas précisé si cette obligation s'appliquerait seulement lorsque les personnes concernées envisagent de stationner sur un terrain public, ou si elle s'appliquerait aussi en cas de stationnement sur un terrain privé, qui pourrait même appartenir l'avis du Gouvernement ?

l'avis de la commission ? Le présent amendement tend à accorder au maire, s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même l'ordre public à l'occasion du stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles dans sa commune, la faculté de demander au préfet de département de prendre les mesures nécessaires. Dans sa version initiale, l'article 3 de la proposition de loi prévoyait de transférer de plein droit au préfet le pouvoir de police générale du maire lors des grands passages et grands rassemblements de gens du voyage. M. Jean-Claude Carle a entendu les réticences exprimées par votre commission à l'idée de ce transfert, lequel aurait privé les maires de toute possibilité légale d'agir pour maintenir l'ordre public lors de ces événements, et il propose ici un dispositif différent. Il convient de rappeler qu'en l'état actuel du droit le préfet dispose de la faculté de se substituer, après mise en demeure, à un maire qui refuserait de prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public dans sa commune. Le préfet agit alors en lieu et place du maire, et il engage la responsabilité de la commune en cas de faute, même simple, dans l'exercice de ce pouvoir de police municipale. En outre, en cas de trouble grave à l'ordre public et face à la carence du maire, si le préfet ne fait pas usage de son pouvoir de substitution, il est susceptible d'engager la responsabilité de l'État pour faute lourde. Le présent amendement envisage une hypothèse différente, selon laquelle le maire ne refuse pas d'agir, mais se trouve dans l'impossibilité matérielle de le faire. Il pourrait alors demander au préfet de prendre les mesures nécessaires. Le préfet conserverait cependant la faculté de rejeter la demande et de laisser au maire le soin d'assurer l'ordre public, quitte à se substituer à lui en cas de carence,

Premièrement, en cas d'acceptation par le préfet de la demande du maire, il semble résulter de la rédaction proposée que le préfet agirait au nom de l'État. Toute faute commise dans l'exercice de ses pouvoirs engagerait donc la responsabilité de l'État. Toutefois, le maire conserverait-il la possibilité légale d'agir ? La commune serait-elle déchargée de toute responsabilité en cas de dommages liés à un trouble à l'ordre public ou à l'exercice des pouvoirs de police ? Deuxièmement, en cas de refus du préfet, celui-ci devrait-il être motivé ? ? Un refus injustifié engagerait-il la responsabilité de l'État ? Cet amendement pose donc des questions qui méritent plus ample réflexion afin, notamment, de lever toute incertitude sur la répartition des responsabilités entre la commune et l'État. Aussi, pour l'heure, je m'en remets à la sagesse du Sénat et je demande l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement ? qui prévoit que « le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages confie déjà la police des rassemblements et des grands passages des gens du voyage à l'État, et ce quel que soit le régime de police dont relève la commune. C'est pourquoi le Gouvernement considère que le droit permet déjà ce que vous proposez.

que le redevable devra apposer de manière visible sur son véhicule. ? La quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a instauré une taxe sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal. Cette taxe revêt la forme d'un droit de timbre, inspiré de l'ancienne vignette automobile, que les propriétaires doivent acquitter chaque année. Cette taxe relève de la procédure de paiement sur déclaration : le propriétaire d'une résidence mobile occupée à titre d'habitat principal doit en faire la déclaration auprès du centre des finances publiques et s'acquitter immédiatement de la taxe due. Un récépissé lui est délivré. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et les EPCI au prorata de leurs dépenses engagées pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'aires et de terrains d'accueil destinés aux gens du voyage. Le présent amendement tend à augmenter le montant de la taxe, en le portant de 150 à 200 euros par an, de 100 à 150 euros pour les résidences mobiles vieilles de plus de dix ans. Il prévoit aussi que le récépissé est délivré par l'administration fiscale sous forme d'une vignette, celle-ci devant obligatoirement être apposée sur le véhicule. Je ne suis pas certaine que cette dernière disposition- la « vignette » -soit de nature à faciliter le recouvrement de la taxe ou la sanction de son non-paiement. On peut d'ailleurs s'interroger sur les modalités de contrôle de cette taxe : lors d'un contrôle routier, si le conducteur du véhicule n'est pas en mesure de produire le récépissé délivré par l'administration, comment l'agent de police ou de gendarmerie peut-il s'assurer que le véhicule est bien utilisé en tant qu'habitation principale ? Le Gouvernement nous éclairera peut-être sur ce point. Il n'en demeure pas moins que l'augmentation du produit de la taxe fournirait aux communes et EPCI des moyens précieux pour construire les aires et terrains d'accueil prévus par les schémas départementaux,

des aires d'accueil des gens du voyage. Cette mesure, qui est de nature à apporter une obole supplémentaire pour mieux gérer ces aides, n'est pas du tout excessive. Au contraire, elle permettra aux communes d'être encore plus performantes dans la gestion de ces aires.

? Cet amendement tend à supprimer la disposition selon laquelle le maire d'une commune dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental dispose du pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune,

Je l'ai déjà indiqué dans mon propos liminaire, le Gouvernement demeure bien sûr attaché à ce que la solidarité au sein de l'EPCI soit le moteur permettant la réalisation de l'ensemble des aires d'accueil prévues au schéma départemental. Pour autant, je suis sensible à la situation un peu délicate des communes qui disposent d'une aire d'accueil, mais qui sont situées dans un EPCI ne remplissant ses obligations. Je peux entendre l'incompréhension des élus de terrain ; c'est absolument évident. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

sauf les aires permanentes d'accueil, les aires de grand passage et les terrains familiaux situés sur le territoire de la collectivité. Cette mesure apparaît disproportionnée, au regard de la notion de liberté d'aller et venir. Le trouble à l'ordre public justifiant l'évacuation s'apprécie au niveau du terrain et non à l'échelle du territoire de la commune ou de l'EPCI. Par ailleurs, cet article modifie l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 pour considérer le trouble à l'ordre public comme une condition possible mais non nécessaire à l'intervention du préfet dans le cadre de la procédure de mise en demeure et d'évacuation. Une telle disposition ne peut être acceptée. En effet, ce n'est que pour garantir l'ordre public que le préfet peut faire usage de ses pouvoirs de police en la matière, comme l'a rappelé récemment le Conseil constitutionnel. De plus, l'article 5 prévoit que que le délai d'exécution de la mise en demeure est de vingt-quatre heures systématiquement si les occupants ont déjà occupé précédemment de façon illicite un terrain sur le territoire de la commune ou de l'EPCI concerné. Or la mise en demeure étant une mesure de police administrative et non une sanction, il n'est pas possible de corréler le délai d'exécution de l'évacuation au comportement passé des occupants du terrain. La différence de traitement opérée entre « récidivistes » ou non méconnaîtrait le principe d'égalité. Qui plus est, les conditions pratiques de mise en oeuvre d'un dispositif- base de données -permettant de constater la réitération et la présence des mêmes personnes semblent complexes. Enfin, l'article vise à établir dans la loi que la condition d'urgence n'est pas requise ou est présumée remplie, en cas d'occupation illégale d'un terrain par des gens du voyage, dans le cadre des procédures d'expulsion pouvant être diligentées devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Une telle présomption d'urgence, appliquée aux seuls gens du voyage occupant illicitement un terrain, encourrait le double grief d'atteinte au principe d'égalité et de discrimination. Quel est l'avis de la commission ? La multiplication des installations « sauvages » justifie de renforcer les procédures existantes, qu'il s'agisse de procédures de police administrative ou de procédures judiciaires. Les arguments avancés par le Gouvernement- veuillez m'en excuser, madame la ministre ! -ne sont pas convaincants. Premièrement, étendre le périmètre de la mise en demeure d'évacuer à l'ensemble de la commune ou de l'EPCI serait « manifestement disproportionné au regard de la liberté d'aller et venir le trouble à l'ordre public s'appréciant à l'échelle de chaque terrain. Pourtant, le droit en vigueur prévoit d'ores et déjà que la mise en demeure du préfet reste applicable ... Absolument ! ... si la même résidence mobile se retrouve de nouveau, dans un délai de sept jours, en stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Le texte de la commission, sur ce point, ne change rien au droit positif : il ne fait que préciser la rédaction de la loi. Deuxièmement, au motif que la mise en demeure est une mesure de police administrative et non une sanction, il ne serait pas possible de différencier son délai d'exécution en fonction du comportement passé des occupants, et de le limiter à vingt-quatre heures en cas de réitération au cours de la même année. La commission des lois est sensible à la nécessité de maintenir une frontière nette entre police administrative et répression pénale. il arrive d'ores et déjà que des mesures de police administrative soient motivées par le comportement passé des personnes. Il en va ainsi de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre d'un étranger, qui prend acte de son comportement passé pour en déduire un risque de trouble à l'ordre public qu'il est nécessaire de prévenir. Troisièmement, l'augmentation de sept à quinze jours de la durée d'applicabilité de la mise en demeure serait « excessive ». En réalité, la durée actuelle de sept jours est nettement insuffisante. Compte tenu des délais incompressibles dans lesquels est enfermée la procédure, il peut s'écouler près d'une semaine entre la mise en demeure du préfet et l'évacuation effective des terrains. Si l'on veut empêcher que des campements illicites ne se reconstituent immédiatement à proximité, il est nécessaire de porter à quinze jours le délai d'applicabilité de la mise en demeure. Quatrièmement, contrairement à ce que l'on peut lire dans l'objet de l'amendement du Gouvernement, le texte de la commission ne limite nullement à quarante-huit heures le délai d'exécution de la mise en demeure.

Cinquièmement, les dispositions introduites par la commission selon lesquelles la condition d'urgence est écartée ou présumée remplie en cas de référé administratif, de référé civil ou de requête civile portant sur l'occupation sans titre d'un terrain par des résidences mobiles seraient attentatoires au principe d'égalité et discriminatoires. de rappeler au Gouvernement que la loi du 5 juillet 2000 prévoit déjà des procédures exorbitantes du droit commun en cas de stationnement illicite de résidences mobiles- la procédure d'évacuation d'office et la procédure civile spéciale en cas d'occupation d'un terrain affecté à une activité économique. Ces procédures sont la contrepartie des droits reconnus aux gens du voyage par cette même loi et des obligations d'accueil faites aux communes et à leurs groupements. Or, à

constatés de nombreux stationnements illicites, qui donnent lieu à une mise en demeure administrative de quitter les lieux. Effectivement, comme on le dit, les gendarmes ou les policiers poussent les gens du voyage en infraction à quitter le terrain en question, ceux-ci vont dans la même commune sur un autre terrain, sur un autre tènement cadastral où ils s'installent de nouveau ou bien ils changent de commune, mais restent dans le même EPCI. Il s'agit d'une question extrêmement concrète

nous sommes dans une période de lutte contre le terrorisme : l'été, la plupart des forces mobiles de police ou de gendarmerie sont occupées à d'autres fonctions que la fonction de

Il modifie la procédure administrative d'évacuation d'office et prévoit d'assouplir les procédures du référé administratif, du référé civil et de la requête civile. La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a déjà renforcé la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée. Elle a également pris en considération le cas d'occupation de terrains affectés à une activité économique parmi lesquels figurent les terrains agricoles, lorsque cette occupation est de est de nature à entraver ladite activité. Ainsi, le droit en vigueur offre déjà toute une palette d'interventions. Indépendamment de la procédure spéciale d'évacuation d'office et de la procédure civile spéciale applicable au stationnement illicite de résidences mobiles sur un terrain affecté à une activité économique, le maire de toute commune conserve la possibilité de faire évacuer d'office un campement sur le fondement de son pouvoir de police générale, en cas de risque grave pour l'ordre public et si l'urgence le justifie. En outre, ces possibilités d'évacuation d'office coexistent avec les procédures juridictionnelles administratives et civiles d'expulsion de droit commun ainsi qu'avec la procédure pénale. Certes, le législateur peut toujours s'employer à rechercher les voies et moyens pour rendre les procédures plus opérantes et plus rapides. Mais est-ce bien fondé quand cette démarche hypothétique revient à défaire une réforme qui a moins d'un an d'existence et qui n'a pu déployer la totalité de ses effets en raison de l'absence de publication de publication des décrets d'application ? Surtout, est-ce réaliste lorsque l'ensemble des observateurs et notre rapporteur conviennent que les difficultés pour faire évacuer les campements illicites tiennent moins à la nature des procédures existantes qu'à l'insuffisance des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ? Vous reconnaissez vous-même que « les préfets ne mobilisent qu'avec parcimonie la force publique pour faire évacuer d'office des campements ou faire exécuter une décision de justice, à l'heure où policiers et gendarmes sont fortement sollicités sur d'autres terrains Ainsi, la limitation à quarante-huit heures du délai de recours contre la mise en demeure d'évacuer les lieux délivrée par le préfet ne changera rien, comme il serait illusoire de croire qu'il suffit de porter de sept à quinze jours la durée d'applicabilité de la mise en demeure en cas de nouveau stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou du même EPCI

au cours de l'année écoulée, car cette mesure n'est assortie d'aucune sanction en cas de défaut d'intervention de la force publique. Vous pouvez donc toujours en exprimer le souhait et même l'écrire, assouplir les procédures du référé administratif, du référé civil et de la requête civile, cela n'en fera pas une disposition législative effective pour autant. L'amendement n° 6 rectifié, Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement tend à modifier le périmètre d'application du maintien de la mise en demeure du préfet prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. En effet, à ce jour, ce dispositif vise uniquement le territoire de la commune ou de l'intercommunalité concernée par le stationnement illicite. Or cette mesure n'est pas adaptée au regard de la situation et ne prend pas en compte la réalité du terrain. Il y a quelques jours, j'étais encore maire et présidente d'une communauté de communes, et, comme beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, j'ai été confrontée à ce problème majeur. Aujourd'hui- c'est notamment vrai dans l'Essonne -, une fois l'ordre donné de quitter les lieux, on observe régulièrement un déplacement de ces installations sur des communes voisines. Aussi, je tiens à souligner que les collectivités territoriales, pour la plupart d'entre elles, ont fait des efforts considérables dans la construction d'aires d'accueil pour les gens du voyage, ... Absolument ! ... Tout au moins, c'est le cas dans le sud de l'Essonne. D'ailleurs, il faut préciser qu'elles ont investi énormément d'argent pour se doter de structures modernes et être, par conséquent, en conformité avec la loi et les schémas départementaux. Dans ces conditions, on ne peut pas accepter de telles occupations illicites. En outre, je puis vous assurer, madame la ministre, mes chers collègues, que cet amendement est à la hauteur de l'exaspération, pour ne pas dire de la colère des élus locaux, qui n'en peuvent plus de subir fréquemment de telles occupations illicites. Ces derniers attendent des solutions concrètes. Il est donc indispensable d'améliorer cette mesure en élargissant l'échelon territorial actuellement visé dans la loi, afin d'éviter l'engagement de nouvelles procédures auprès du préfet et de mieux lutter contre ces agissements qui, je vous l'assure, épuisent les maires. Enfin, cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de cette proposition de loi, à savoir plus de clarté et de justice pour nos territoires. Voilà pourquoi je propose d'étendre les effets de cette mise en demeure au niveau départemental. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement ? L'amendement n° 23 tend à supprimer la plus grande partie de l'article 5 relatif au renforcement des procédures d'évacuation des résidences mobiles irrégulièrement stationnées. Il est vrai que les difficultés rencontrées sur le terrain tiennent avant tout à l'insuffisance des moyens dont disposent les préfectures pour faire évacuer les campements, d'office ou en exécution d'une décision de justice. Policiers et gendarmes sont, aujourd'hui, fortement sollicités sur d'autres terrains. Il n'en reste pas moins que les procédures elles-mêmes méritent d'être précisées et renforcées. À titre d'exemple, dans le cadre de la procédure administrative d'évacuation d'office, aucun délai de recours contre la mise en demeure du préfet n'est actuellement prévu par la loi. Il semble parfaitement légitime de limiter ce délai de recours à quarante-huit

Elle s'est attachée à faciliter le recours à la procédure sur requête, une procédure non contradictoire admise par le juge lorsqu'il est impossible d'assigner en justice l'auteur d'un trouble dont on demande la cessation. En conséquence,

Cet amendement concerne le périmètre d'application de la mise en demeure du préfet : la mise en demeure resterait applicable dans un délai de quinze jours, comme le prévoit la proposition de loi, si la résidence mobile concernée se retrouvait de nouveau en stationnement illicite, en violation du même du même arrêté, sur le territoire du département, et non plus seulement sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Cette proposition se heurte à une impossibilité juridique, puisque l'arrêté dont il est question est un arrêté du maire ou du président de l'EPCI compétent, applicable sur le territoire de la commune ou de l'EPCI, et pas au-delà. C'est la violation de son arrêté qui permet au maire ou au président de l'EPCI de saisir le préfet et de mettre ainsi en mouvement la procédure d'évacuation d'office. Si les contrevenants se retrouvent de nouveau, dans un délai de quinze jours, en stationnement illicite sur le territoire d'une autre intercommunalité, c'est nécessairement en violation d'un autre arrêté, et cela nécessite que le maire ou le président de l'EPCI concerné prenne à son tour l'initiative d'une demande au préfet de mise en demeure. En outre, le périmètre proposé, qui couvrirait l'ensemble du territoire départemental, paraît excessif. Un nouveau stationnement irrégulier dans un autre EPCI, en violation d'un autre arrêté municipal ou intercommunal, constitue un trouble à l'ordre public distinct, qui justifie qu'une nouvelle mise en demeure soit adressée par le préfet avant l'évacuation forcée. Enfin, l'amendement n'aurait qu'une portée pratique limitée. Certes, la seconde mise en demeure est assortie d'un nouveau délai d'exécution, mais celui-ci peut être limité à vingt-quatre heures. Compte tenu de la difficulté rencontrée par les préfectures à mobiliser les forces de l'ordre pour de telles opérations, la mesure proposée permettrait, tout au plus, d'évacuer les campements illicites quelques

n° 23. Concernant l'amendement n° 6 rectifié, je reprendrai l'argumentation au fond de Mme le rapporteur. Comme pour toute mesure de police administrative, la validité juridique du dispositif de la mise en demeure n'est garantie que si elle est adaptée et proportionnée au but visé. Dans une décision en date du 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a rappelé que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif. Dans le cas présent, l'extension de l'applicabilité de la mise en demeure aux autres communes du département département est manifestement excessive. Cette mise en demeure intervient notamment en cas de violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public.

Il double les peines prévues à l'article 322-4-1 du code pénal, avec une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 7 500 euros. En outre, il applique à cette infraction la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle fixée à 500 euros, 400 euros lorsqu'elle est minorée et 1 000 euros lorsqu'elle est majorée. Enfin, il supprime la protection accordée aux véhicules destinés à l'habitation contre les saisies et confiscation. Le doublement des peines proposé à l'article 6 ne permettra pas de mieux prévenir les occupations illicites de terrains puisque les sanctions en vigueur s'avèrent déjà faiblement prononcées par les juges. Se poserait de plus un problème de nécessité et de proportionnalité. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle sera inopérante dès lors qu'elle s'appliquera pour sanctionner l'infraction d'occupation illicite en réunion et non individuelle. Il en est de même de l'assouplissement des conditions de saisie et de confiscation des véhicules, en raison des frais de justice liés tant à l'évacuation qu'au gardiennage qu'il faudra engager et des capacités réduites de mobilisation des forces de l'ordre sur ces questions. Enfin, la faculté de saisir des véhicules destinés à l'habitation ne respecte probablement pas l'équilibre nécessaire entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie liée à l'inviolabilité du domicile. Quel est l'avis de la commission ?

Certes, le délit n'est constitué qu'à partir de deux caravanes ; mais cela n'empêche nullement de dresser des procès-verbaux pour chaque caravane qui participe à l'infraction. En effet, chaque participant individuel à l'infraction est susceptible d'être condamné pour ce délit ou de faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. Les auteurs du présent amendement considèrent que la saisie des véhicules destinés à l'habitation n'est pas équilibrée. Je rappelle que le code pénal et le code de procédure pénale permettent déjà de saisir des domiciles. Tout bien susceptible d'être confisqué peut être saisi et, en application d'une disposition générale du code pénal, tout bien ayant servi à commettre une infraction peut être confisqué. Or il est évident que les résidences mobiles, en cas d'occupation illicite, participent à la commission d'une infraction. La suppression de la protection accordée aux véhicules d'habitation n'est pas dérogatoire ; elle permet simplement de revenir à l'application normale des règles en matière de saisie et de confiscation. je rappelle que, pour un certain nombre de délits, la confiscation peut porter sur tout bien appartenant au patrimoine du délinquant. Dans ces cas-là, le lieu d'habitation peut être saisi, puis confisqué. Certes, la confiscation du domicile constitue une atteinte au droit de propriété- davantage qu'à l'inviolabilité du domicile, dont la protection est inopérante s'agissant d'une décision juridictionnelle contradictoire

objet si cet amendement était adopté. Plutôt que de faire de l'installation illicite un motif d'aggravation de la dégradation d'un bien appartenant à autrui, nous proposons de faire de la dégradation d'un bien appartenant à autrui une circonstance aggravante de l'installation illicite, ce qui paraît plus logique.

autrui. Quel est l'avis de la commission ? d'aggraver les sanctions applicables au délit d'occupation illicite quand celui-ci s'accompagne de destructions, détériorations ou dégradations d'un bien d'autrui et, en conséquence, de supprimer la circonstance aggravante prévue à l'article 7 du texte de la commission. Cette proposition de M. Patriat aurait pu être un choix pertinent, mais elle présente un inconvénient majeur : elle ne permet pas d'aggraver les peines en cas de commission de deux Or le dispositif répressif des destructions, détériorations ou dégradations d'un bien d'autrui est construit de manière graduée dans le code pénal : il permet des sanctions de plus en plus fortes en cas de circonstance aggravante, voire de pluralité de circonstances aggravantes. Les peines peuvent être portées jusqu'à sept ans d'emprisonnement si deux circonstances aggravantes sont réunies : par exemple, lorsqu'une dégradation a été commise au cours d'une occupation illicite et que le bien dégradé est destiné à l'utilité publique et appartient à une personne publique.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'installation est précédée, accompagnée ou suivie de l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1.

En effet, la saisie et la confiscation de véhicule ne peuvent concerner un véhicule servant de lieu d'habitation. Une telle mesure, qui aurait pour effet de priver de toit l'auteur des faits, contrevient au principe de l'inviolabilité du domicile qui est protégé constitutionnellement.

Le présent amendement vise à supprimer également la possibilité donnée au juge de transférer les véhicules sur une aire ou un terrain d'accueil situé sur le territoire du département. cette disposition ne paraît pas conforme au principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi : elle est insuffisamment précise, dans la mesure où elle ne prévoit pas les modalités de son application. au surplus, s'annonce délicate sur le plan opérationnel, s'agissant d'une mesure innovante en matière pénale de déplacement d'un objet appartenant à autrui, qui s'apparente à une saisie. En outre, cette mesure appelle les mêmes remarques qu'en matière de saisie concernant les véhicules destinés à l'habitation et porte atteinte au principe d'inviolabilité du domicile.

Avec l'article 6, nous entamons l'examen du chapitre III de la proposition de loi qui renforce les sanctions pénales et le dispositif répressif. Ce chapitre, disons-le d'emblée, est celui qui nous laisse le plus circonspects. L'alinéa 6 de l'article 6 rend possible la saisie des véhicules d'habitation en cas d'installation illicite. Mme la ministre nous a fait part de ses réserves quant à la conformité d'une telle mesure avec les grands principes constitutionnels. Celle-ci semble en effet contrevenir au principe d'inviolabilité du domicile.

Pour être concret, imagine-t-on les forces de l'ordre procéder à la saisie des caravanes des gens du voyage, alors même que ces dernières sont leur résidence principale ? J'ai été maire et j'ai vu mon terrain de camping envahi ... Je vois mal comment on pourrait saisir des caravanes

au cours d'une installation illégale d'un groupe de gens du voyage pourrait sembler une disposition de bon sens. En effet, pourquoi ne pas trouver les voies d'une sanction plus forte dans les cas où l'occupation illégale d'un terrain se double de dégradations ? Il apparaît toutefois que les condamnations au titre de l'article 322-4-1 du code pénal sont à ce jour particulièrement peu nombreuses. Il y a donc fort à parier qu'une telle évolution législative n'améliorerait en rien la situation que connaissent les maires et certains de nos concitoyens sur le terrain. Alors que l'objet affiché est de rendre les sanctions plus effectives, je crains pour ma part que cet article ne les rende que plus virtuelles

La question à laquelle sont confrontées les autorités publiques est de répondre concrètement aux difficultés qui se posent sur le terrain, non d'afficher des postures sans efficacité ! Quel est l'avis de la commission ?

Permettra-t-elle une évacuation plus rapide des occupations illicites ? Aura-t-elle des vertus dissuasives ? On peut en douter ! Je pense qu'inscrire dans le code pénal des délits et des sanctions afférentes tout en sachant très bien que celles-ci ne peuvent s'appliquer

en réunion sans titre sur le terrain d'autrui prévu à l'article 322-4-1 du code pénal. Or cette disposition est inapplicable, car l'article 495-17 du code de procédure pénale, qui régit la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, prévoit, dans son second alinéa, que cette procédure n'est pas applicable si le délit a été commis en état de récidive légale. La récidive étant appréciée sur une période de cinq ans, selon l'article 132-10 du code pénal, l'auteur du délit prévu à l'article 322-4-1 du même code ne peut se voir appliquer la procédure de l'amende forfaitaire qu'une seule fois durant une période de Le délit d'occupation habituelle ne trouvera donc pas à s'appliquer. En conséquence, le Gouvernement propose de supprimer l'article 8 de la proposition de loi. Quel est l'avis de la commission ? La commission

et en réunion d'un terrain. Ce type de délit a démontré son efficacité en matière de lutte contre les transports, où un délit similaire de fraude habituelle existe. La création de ce délit complète utilement l'arsenal pénal

: elle considère que, en l'état actuel du droit et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la récidive légale ne se constate qu'en cas de réitération d'une infraction après une condamnation devenue définitive, qui suppose une déclaration de culpabilité par une juridiction de jugement après mise en mouvement de l'action publique. Or une amende forfaitaire délictuelle, au même titre qu'une amende de composition pénale, par exemple, n'est pas une condamnation

au regard de la peine principale encourue en cas de délit d'installation illicite, même si celle-ci a été portée à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende par l'article 6 de la présente proposition de loi. vise également à rétablir l'exclusion de la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction quand il s'agit d'un véhicule destiné à l'habitation, car cette confiscation serait

exemple applicable en cas de délit de demande de fonds sous contrainte qui est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement. Ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003. La peine complémentaire d'interdiction de séjour est également applicable au délit prévu à l'article 431-22 du code pénal, qui réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans autorisation. Ce délit et les peines complémentaires afférentes créés par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public ont également été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 février 2010. En conséquence, l'application de cette peine complémentaire à des infractions punies d'un an d'emprisonnement n'est pas disproportionnée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

et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n° 21,